Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Bruno Le Maire, ministre des Finances et des Comptes publics.

Monsieur le président. J'allais dire, monsieur le rapporteur général mais vous transmettrez. Au rapporteur général Albéric de Montgolfier tous mes souhaits de prompt rétablissement puisque je comprends qu'il a dû. être hospitalisé en urgence, ce matin, monsieur le ministre, chers Gérald mesdames et messieurs les sénateurs. Ce projet de loi de finances pour 2018 le 1er du nouveau quinquennat. Il traduit la vision économique porté par le gouvernement. Il s'inscrit dans une stratégie globale clairement annoncé par le président de la République pendant sa campagne et choisi par les Français. Transformer le modèle économique de notre pays. Pour cela, parce qu'on aborde la situation économique. International. La reprise mondiale se confirme avec une croissance globale qui est estimé à 3,6 pourcent pour 2017 dans le monde. Les prévisions les plus récentes, notamment celle du FMI annonce un rythme équivalent pour 2018. Le continent européen se place et cela mérite d'être noté dans le peloton de tête. La reprise économique se poursuit à un rythme solide dans la zone Euro. La croissance économique dans l'Union monétaire devrait être de 2 pourcent en moyenne cette année. En France, les principaux indicateurs économiques se redresse. En un an 300000 emplois ont été créés dans le secteur marchand. L'investissement retrouvent un rythme soutenu. La création d'entreprise également, la confiance est donc de retour chez les entrepreneurs. Et j'estime que la croissance française est désormais une croissance solide. Dans cette conjoncture favorable, nous voulons accélérer la transformation économique de la France. Nous voulons éviter de reproduire les erreurs qui ont été trop souvent commises ou à la moindre amélioration de la conjoncture, on reportait les transformations économiques nécessaires, nous nous estimons au contraire que parce que les choses vont mieux. Il faut accélérer la transformation économique du pays pour qu'il puisse exploiter à plein, c'est talent et ses atouts qui sont eux immense. La réforme du marché du travail, le budget que nous discutons aujourd'hui la raison. Forme de la formation professionnelle et demain de l'assurance chômage marque notre détermination dans cette majorité à accomplir la transformation économique et sociale du pays, sous l'autorité du président de la République. Sous l'autorité du 1er ministre nous irons jusqu'au bout dans cette transformation nécessaire. Le monde. Ne nous attendra pas. Les autres nations ne nous attendront pas. Les grandes puissances comme la Chine ou comme les États-Unis, ne nous attendront pas. Si nous voulons rester une puissance économique de 1er plan. Nous devons saisir les révolutions technologiques en cours. Faute de quoi nous serons rejetés dans les marges appauvri. Nos choix économiques ont un but clair : permettre à la France de répondre aux défis contemporains et de réussir dans le monde, telle qu'il est. Pour cela, la première exigence et de permettre à nos entreprises d'investir. Et pour investir, encore faut-il qu'elle retrouve la profitabilité. C'est pour cela qu'une des décisions majeures que nous vous proposons avec Gérald Darmanin c'est de l'allégement de la fiscalité sur le capital. Alléger la fiscalité sur le capital, c'est renforcer la profitabilité de l'entreprise qui est trop faible, et c'est leur permettent d'investir pour innover. Les solutions du passé ont eux échoué. Les solutions consistant à redistribuer de la richesse avant de la créer ont échoué. Nous vous proposons une autre voie. Celle qui consiste à alléger la fiscalité sur le capital pour dégager les moyens nécessaires à nos entreprises pour qu'elles investissent pour qu'elles innovent. Pour qu'elle reste en tête la course technologique actuelle, regardez les taux marginaux d'imposition actuelle sur le capital

Comment voulez-vous que nous entrepreneurs. Puisse faire la course en tête quand ils ont un pareil boulet au pied, nous allons alléger la fiscalité sur la capitale pour récompenser le risque pour faciliter l'investissement pour faciliter le financement de nos entreprises, sans capital, pas d'investissement sans investissement, pas d'innovation sans innovation, pas d'emploi. Nous voulons rompre avec cette fâcheuse habitude française. De redistribuer les richesses, avant de les avoir créées parce qu'au bout du compte, cela affaiblit tous les Français. Et cela affaiblit la souveraineté de la France. Alléger cette fiscalité sur le capital. Cela passe par une décision historique. La mise en place d'un prélèvement forfaitaire unique à 30 pourcent. Surtout, les revenus du capital. Ce sera un gage de simplicité, ce sera également un gage de meilleure de financement de notre économie. 80 pourcent des pays européens ont déjà adopté une fiscalité proportionnelle de ce type. Mais nous avons aussi été attentif. à ne pas pénaliser la fiscalité de l'épargne salariale pour marquer notre volonté de récompenser le travail, le travail et capital doivent plus être opposé, travail et capital. Doivent aller de Pair. Il faut alléger la taxation du capital pour ne pas le faire fuir dans un monde où le capital est de plus en plus mobiles mais il faut aussi. Redonner sa valeur au travail. Il faut que toutes les Françaises et tous les Français qui vont travailler. Qui ont des niveaux de rémunération parfois faibles. Puis, se dire qu'en travaillant, ils auront la récompense de leurs efforts. Nous voulons maintenir les avantages des produits d'épargne populaire Livret A Livret développement durable resteront entièrement défiscalisé pour les ménages français, nous maintiendrons les avantages des produits fortement investis en actions, comme le PEA, par souci de cohérence avec le besoin de financement de l'autre, économie. Pour la fiscalité de l'assurance-vie qui a suscité tellement de débat dans cet hémicycle et à l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les revenus des futurs versements seront concernés, donc nous ne prenons personne par surprise, je rappelle que ne seront concernées que les assurances vie avec un encours supérieur à 150000 euros, c'est-à-dire des gens courent très élevés pour les encours inférieurs. La fiscalité ne change pas, et je rappelle que ces encours représentent 94 pourcent. Il est essentiel également de rappeler que le P. fut demeure une option et que les contribuables qui veulent faire le choix de rester au barème pourront le faire, si cela est plus intéressant pour eux. Pour faciliter l'accès au capital des entreprises. Pour redonner à nos entrepreneurs et à l'ensemble de notre économie les moyens de mieux se financer. Nous supprimons l'impôt sur la fortune. Pourquoi cette suppression. Parce qu'il faut réinjecter des capitaux. Dans l'économie française. Parce qu'il faut attirer les investisseurs. Nous avons besoin pour développer nos entreprises pour les renforcer pour créer des emplois en France pour enrayer la fuite des talents pour récompenser le risque hein. Arrêtons avec l'idéologie. Regardons ce qui est bon pour le pays, bon pour les entrepreneurs, bon pour la création de richesses, bon pour l'emploi, bon pour la valorisation de risques, bon pour la récompense du travail. Et respecteront ces valeurs, ce serait une manière de respecter le travail des Françaises et des Français et de respecter le goût du risque de nous entrepreneurs, le capital, j'ai dit tout à l'heure et de plus en plus mobiles. Est ce que nous voulons qu'il parte ou est-ce que nous voulons qu'il reste est-ce que nous voulons qu'il aille s'investir à l'étranger ou est-ce que nous voulons qu'il aille s'investir dans nos entreprises françaises pour qu'elles puissent enfin grandir pourquoi notre tissu de PME, dont chacun sait et vous connaissez les territoires ici mieux que personne, chacun sait que notre tissu de PME et trop fragile que ces PME sont trop petites, qu'elles dépendent trop de la dette parce qu'elles n'ont pas assez de fonds propres et bien redonnant du capital ces entrepreneurs nous leur permettrons de grandir, d'affronter la concurrence d'investir et de se projeter sur les marchés extérieurs, où se trouve la croissance et les emplois pour les Français. Pourquoi maintenir hein. Un impôt sur la fortune immobilière tout en supprimant l'ISF. Tout simplement parce que un Euro investi dans l'immobilier notamment ancien ne crée pas le même effet d'entraînement qu'un Euro investi dans une entreprise, je rappelle que cet impôt sur la fortune immobilière ne fera aucun perdant. Je rappelle qu'il reprend exactement les mêmes règles que l'ISF sur le volet immobilier même seuil même abattement de 30 pourcent sa résidence principale, il y a tout ce qu'il me disent. Que nous allons affaiblir la classe moyenne, que nous n'avons pas la même conception de certains, la classe moyenne, puisque je rappelle que l'impôt sa fortune immobilière ne concernera que les biens immobiliers de plus d'1,3 millions d'euros, avec un abattement de 30 pourcent c'est-à-dire un bien immobilier d'un virgule 7 millions d'euros. Le secteur du logement par ailleurs bénéficie déjà d'un certain nombre de dispositifs favorables avec des incitations fiscales puissantes comme l'exonération de la plus-Value sur la vente de la résidence principale ou le prête au 0 et le dispositif Pinel, que nous allons pérenniser. Est-ce pour autant que notre modèle social va devenir inégalitaire. Car j'entends cette critique qui a été faite. Depuis le début des débats sur le PLF pour 2018 critique que nous entendons avec Gérald Darmanin on nous dit : voilà vous libérer des capitaux pour les entrepreneurs ou ou supprimer l'ISF, vous mettez en place le prélèvement forfaitaire unique vous alléger l'impôt sur les sociétés, mais dans le fond. Vous allez créer davantage d'inégalités que d'égalité, je crois, exactement le contraire. Je refuse ces caricatures du budget que nous portons avec Gérald Darmanin je n'accepte pas cette critique. Que le budget du président de la République du 1er ministre de l'ensemble du gouvernement serait un budget pour les riches, c'est un budget pour les Français, c'est un budget pour le travail, c'est un budget pour l'emploi parce que les décisions fiscales que nous prenons permettront enfin, à nous entrepreneurs, de créer des emplois. De créer des richesses pour les Français ont tellement besoin, la première, les inégalités. C'est le chômage. Et la meilleure façon de lutter contre le chômage. C'est de donner à notre économie. Les moyens de mieux se financer. De donner à nos entrepreneurs la récompense de leurs risques. Et de donner à tous ceux qui travaillent la récompense de leurs efforts, voilà la philosophie politique qui nous anime, derrière ce projet de budget pour 2018 la récompense de l'effort, la récompense des salariés, la récompense du travail, la valorisation du risque, le soutien à nos entrepreneurs, la capacité à mieux financer l'indépendance et la souveraineté financière d'une nation qui arrête de trop taxé et qui se donne les moyens de créer les richesses dont elle a besoin.

Je rappelle, par conséquent, que lorsque on vous regardez la question majeure des inégalités dans notre pays, il faut pas uniquement regarder ce qui est fait en matière de fiscalité. Il faut également regarder la redistribution sociale qui était la meilleure façon de lutter contre les inégalités et dont nous maintenons l'architecture principal. Le budget que nous vous présentons comporte également une politique ambitieuse en faveur des entrepreneurs. Nous allons baisser l'impôt sur les sociétés de 33 véhicules 3 pourcent à 25 pourcent d'ici la fin du quinquennat soit plus de 11 milliards d'euros de moins de charges fiscales pour les entreprises. Ce choix est un choix structurants dans le budget. Un choix que nous revendiquons avec Gérald Darmanin. Avec le 1er ministre. Avec le président de la République. Nous estimons que nos entreprises doivent être plus profitable. Et que le taux de marge des entreprises qui n'a cessé de se dégrader depuis des années, qui s'est récemment redressée. Ne s'est pas suffisamment redresser pour leur permettre de dégager les moyens d'investir et de créer de nouvelles richesses. Alléger la fiscalité sur les entreprises, c'est renforcer leur capacité à créer des emplois. Nous commencerons avec un taux de 28 pourcent dès 2018 sur la fraction de bénéfice inférieur à 500000 euros nous baisserons ensuite le taux à 31 pourcent pour tous les bénéfices à partir de 2019 tout en maintenant le taux de 28 pour 100 pour des bénéfices inférieurs à 500000 euros. Ce sera ensuite 28 pourcent en 2020 pour tous les bénéfices 26,5 pourcent en 2020 et 1 et 25 pourcent de taux d'impôts ces sociétés en 2022. C'est le taux d'impôt sur les sociétés les plus faibles en France depuis plusieurs décennies. Nous maintiendrons évidemment le taux réduit de 15 pourcent pour les PME qui en bénéficient déjà, parce que nous avons parfaitement conscience que les PME sont celles qui ont aujourd'hui le plus besoin de notre soutien. Vous me direz que nous avons mis en place une contribution exceptionnelle dans le récent projet de loi de finances rectificative. Qui va à l'inverse de cette politique. Je vais pas rouvrir les débats cette contribution exceptionnelle. Nous avons déjà passé beaucoup de temps mais je ne voudrais pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt. Cette contribution exceptionnelle elle être exceptionnelle, elle n'a pas vocation à être reproduite. Elle est pour 2017, point barre, et ensuite nous retrouvons le cap qui est celui du quinquennat la baisse de l'Inde. Sur les sociétés, la baisse des prélèvements sur les bénéfices et le soutien à nos entreprises, nous supprimerons également le CICE pour le transformer en allégement de charges pérenne. Cet allégement passe de 7 à 6 pourcent en 2019 mais je rappelle qu'en 2019, les entreprises ont bénéficié à la fois de ce CICE à un taux ramené à 6 Et de l'allégement de charges directes, donc elles auront en 2019, un Avantage fiscal considérable. J'ajoute enfin. Que le 1er ministre a souhaité que nous ouvrions la réflexion sur les allégements de charges, au-dessus de 2,5 SMIC. C'est un changement majeur. Car pour la première fois. Depuis plusieurs années. Nous estimons. Que les allégements de charges. Ne doivent pas uniquement répondre au défi de l'emploi. Ils doivent aussi répondre au défi de la compétitivité de notre industrie. Nous avons déjà eu aussi, ces débats dans cet hémicycle, ce sont des débats majeurs oui les allégements de charges sont efficaces sur les bas salaires, pour que les plus fragiles et les moins qualifiées, puissent trouver un emploi et leur place dans la société française. Mais oui, nous devons aussi tenir compte de la situation de notre industrie, il faut pas oublier que nous avons perdu 1,4 1000000 d'emplois en 25 ans dans l'industrie française, nous ne devons pas oublier que notre industrie, notre Patrimoine industriel. Qui représentait 20 pourcent de la richesse nationale, il y a 25 ans ne représentent plus que 13 pourcent aujourd'hui alors à tous ceux qui me dit : il faut continuer comme avant, on ne touche rien, on ne change rien, modifie rien jeudi dans en est hors de question. Le statu quo ne peut pas être une solution pour notre industrie. Nous avons besoin de retrouver en compétitivité, ça passe par une ovation. Mais ça passe aussi par l'allégement des charges ces salaires les plus qualifiés, parce que les salaires les plus qualifiés sont l'avenir de notre industrie. Nous ouvrirons donc cette réflexion et comme l'a indiqué le 1er ministre Édouard Philippe, nous mettrons cela en oeuvre quand la restauration des comptes publics et seulement à ce moment-là, nous le permettra. Nous maintiendrons également les dispositifs de soutien à la recherche, le crédit impôt recherche sera sanctuarisée, parce qu'il fonctionne parce qu'il a apporté la preuve de son efficacité, nous mettrons en place au début de l'année 2018 un fonds pour l'innovation de rupture 10 milliards d'euros financés par des cessions d'actifs de l'État dans le secteur concurrentiel. Parce que l'argent de l'État sera tout de même mieux employé à investir dans l'innovation, de recherche, pour préparer l'avenir de nos enfants plutôt qu'à toucher des dividendes d'entreprises nous ne contrôlons pas suffisamment le fonctionnement. Voilà notre stratégie fiscale. Voilà ce qui doit permettre. à nos entreprises. à notre économie. De réaliser enfin son potentiel qui est considérable. Nous sommes convaincus que ces choix seront efficaces, alors oui. Ce sont des choix de rupture. Oui, ce sont des choix qui aurait dû être fait il y a 10, 20 ou 30 ans et que nous ne faisons quand maintenant. Et parce qu'ils sont nouveaux. Nous sommes prêts à les évaluer. La meilleure réponse aux critiques qui sont toutes légitimes en démocratie, c'est la transparence. C'est l'évaluation. Je suis prêt à engager une évaluation d'ici 2 ans de notre politique fiscale. Nous mettrons en place, comme je l'avais promis. Une mission de suivi qui pourra rendre ses premières conclusions dans 2 ans. Cette mission sera composée de parlementaires. 2 membres de la Cour des comptes. Le représentant de l'administration compétente. Le Trésor l'INSEE. 2 personnalités qualifiées et pourquoi pas ajouter à cette mission des entrepreneurs. Qui pourront aussi participer à cette évaluation de la politique fiscale et juger de ces résultats. Cette mission examinera les effets d'autres réformes sur l'orientation de l'épargne des Français. Sur l'investissement des entreprises sur l'attractivité du territoire sur l'emploi soit inégalités de revenus sur le Patrimoine. Je suis prêt à ce que nous regardions l'ensemble des effets de cette politique fiscale parce que réconcilier les Français. Et l'engagement politique, c'est assumer la transparence cette capable de rendre des comptes et c'est assumer l'évaluation sincère. Honnête de nos politiques publiques. Nous travaillons également avec les institutions bancaires pour qu'elles proposent des produits adaptés à leurs clients. De façon à ce que le capital qui a été libéré, effectivement, s'investir dans nos entreprises et de notre tissu économique, un travail de concertation. Organisée par les députés de la majorité notamment Amélie de Montchalin, il doit permettre de faire évoluer les mentalités et d'orienter l'épargne vers le financement de nos entreprises, c'est au début de l'année que nous aurons les premières propositions sur ce sujet et cette avant le 1er avril 2020, un 1er rapport sera transmis au Parlement sur l'évaluation, la politique fiscale du gouvernement. J'ai lu comme vous. Hier. Les remarques de la Commission européenne. Sur. Mot déficit et. Notre dette. Je veux redire ici. La détermination totale. Du président de la République. Du 1er ministre. L'ensemble du gouvernement. à tenir nos engagements européens. Nous tiendrons nos engagements européens. Nous respecterons les règles de déficit pour 2017. Et nous serons en dessous. La limite des 3 pourcent qui nous a été fixé. Et que nous avons nous-mêmes. Choisi de respecter. La France qui se moque de ses engagements européens. C'est fini. La France qui balaye d'un revers de la main les critiques de ses partenaires européens, c'est fini. La France, qui estime qu'elle peut toute seule. Dicter sa propre conduite. Sans écouter ce que nos partenaires européens ont à nous dire, alors que nous sommes engagés dans le même projet politique, c'est fini. La France, qui ne se soucient pas de bien tenir ses comptes publics, c'est fini, la France qui votent des Budgets qui sont insincère ou les financements nécessaires aux politiques publiques ne se trouve pas inscrit au budget de la nation, c'est fini.

Nous avons dû absorber. En 2017. Nous avons dû absorber en 2017. Nous avons dû absorber en 2017. 8 milliards d'euros de dépenses. Qui n'avait pas été budgétés. Le contentieux de la taxe à 3 pourcent sur les dividendes. Alourdie de 10 milliards d'euros. La charge qui pèse sur les comptes de l'État. C'est un fardeau de 18 milliards d'euros. Il a fallu intégrer à nos comptes. Pour 2017. Voilà la stricte réalité des chiffres. Je ne suis pas là pour juger.

Et nous tiendrons bien les comptes de la nation, oui, il y a un fardeau de 18 milliards d'euros qui pèse aujourd'hui sur l'État français. Et malgré ce fardeau, nous serons en dessous des 3 pourcent de déficit public en 2017, c'est un effort considérable, mais c'est un effort juste et c'est un effort nécessaire. Nos prévisions confirment. Que nous serons en deçà des 3 pourcent de déficit cette année. Permettant à la France. De sortir de la procédure de déficit excessif, où elle est depuis 2009. La Commission européenne a confirmé. Que nous étions en mesure. De sortir en 2018. La procédure pour déficit excessif dans laquelle nous sommes, depuis 2009. c'est une responsabilité collective. Il faut savoir vous tous ici, et nous tous ici, ce que nous voulons pour la France. Je le redis, je ne juge personne, je ne suis pas là pour regarder le passé, je vous dis simplement pour l'avenir. Que souhaitez-vous est-ce que vous souhaitez un budget sincère. C'est ce que nous vous proposons. Est-ce que vous souhaitez, respecter les règles européennes, c'est ce que nouveau proposant est-ce que vous souhaitez que la France sorte oui ou non de la procédure pour déficit public excessif, c'est ce que nous vous proposons et j'espère avoir avec Gérald Darmanin votre soutien sur ces gens ambitions nationales et européennes. Nous avons fait un double choix. eu de tenir les engagements de campagne du président de la République. Et celui de tenir nos engagements européens. Nous avons pris les mesures nécessaires, nous avons donné la sincérité à la loi de finances, nous vous proposons un projet de loi de finances rectificative pour tenir compte de l'aliénation de la taxe à 3 pourcent sur les dividendes. Au-delà de 2017. Nous continuerons à tenir ce cap économique et politique. Avec la baisse des impôts et la maîtrise des dépenses. Car c'est la meilleure façon de renforcer notre croissance potentielle et de réduire le déficit structurel français. Nos obligations européennes nous impose, en effet, au-delà du respect de la règle des 3 pourcent sur le déficit. Pour sortir de la procédure pour déficit excessif de réduire graduellement notre déficit structurel. Et c'est le point sur lequel la Commission européenne s'est arrêté le plus longuement. En 2018, nous prévoyons une réduction de 0 des, de 1 pourcent du déficit structurel. La Commission européenne fait une autre évaluation. Mais il était arrivé dans le passé que les évaluations de la France soit finalement davantage confirmé par les fêtes que celle de la Commission européenne, nous sommes donc en discussion avec la Commission européenne pour faire converger nos chiffres. Nous souhaitons que la Commission prenne en compte la sincérité des mesures qui sont prises dans ce projet de loi de finances, ce qui n'est pas encore le cas et ce qui explique largement les cas entre nos estimations de correction de 0 de 1 pourcent du déficit structurel. Et celle de la commission, qui estime à l'inverse que le des ajustements de 0 virgule 4 points. La Commission doit également prendre en compte l'ensemble des réformes structurelles que nous portons. Et qui vont porter leurs fruits. Réforme de la fiscalité, rationalisation des dépenses qui sera accentuée dès que la revue des dépenses aura permis d'identifier précisément les marges, réforme du code du travail, réforme de l'assurance chômage. Toutes ces mesures structurelles, nous souhaitons que la Commission européenne en prennent davantage compte dans l'évaluation de la réduction de notre déficit structurel j'en parlerai prochainement aux membres de la Commission européenne. En respectant nos engagements européens. Non seulement nous garantissons la bonne tenue des comptes publics de la nation. Mais nous garantissons surtout la restauration de la crédibilité de la parole. La France en Europe. Le président de la République a réussi à obtenir une transformation en profondeur de la directive, ces travailleurs détachés, c'est parce que la France a retrouvé la crédibilité sur la scène européenne. Nous avons relancé le débat sur la taxation des géants du numérique qui est un débat absolument majeur sur l'avenir de la fiscalité internationale, c'est parce que la France. à retrouver sa crédibilité sur la scène internationale. Comment voulez-vous que nous avions expliqué. Aux entrepreneurs de vos territoires, qu'ils soient dans le bâtiment, dans la restauration, dans la chimie, l'industrie automobile. Qu'ils auront à payer leurs taxes locales et leur impôt sur les sociétés, alors que Google Amazone ou Facebook ne paient que des impôts dérisoires au Trésor public français, nous ne lâcherons rien rien rien sur la taxation des géants du numérique. En France et en Europe. Ils lutteront également. Contre le dumping fiscal en Europe. Avec un objectif clair réduire les écarts entre les taux d'imposition européen à la fin du quinquennat. Fr dépendent de cet écart, comme l'a dit le président de la République, le versement des aides européennes pour les fonds structurels, or certains États me disent déjà, mais c'est notre modèle, notre modèle économique, c'est le dumping fiscal. Eh bien, de la même manière qu'on a dit à la France. Que notre modèle de dépenses publiques. On ne pouvait pas être un modèle pour l'Europe, ce qui nous a amenés à faire des efforts. Ce qui m'amène aujourd'hui à vous présenter avec Gérald Darmanin, un budget nous baissons l'impôt sur les sociétés, nous baissons le niveau d'imposition. Nous mettons en place un prélèvement forfaitaire unique. Certes, notre modèle consistant à dépenser plus d'argent et plus de richesses que nous créons n'était pas un modèle qui pouvait être inspirant. Pour les autres États européens. Eh bien, de la même manière, jeudi à tous ceux qui font du dumping fiscal. Le modèle économique de l'Europe, je leur réponds non, ni le dumping fiscal, ni le dumping social ne peuvent être un modèle pour l'avenir de la construction européenne. à chacun de faire des efforts. Nous en faisons. Que nos partenaires en face également c'est uniquement si chacun fait un pas dans la direction de l'autre que l'avenir de l'Europe se construira de manière positive pour tous les citoyens européens. Notre budget tente également. Et transformer notre modèle économique. En faisant bénéficier à tous les Français. Les résultats de cette transformation économique. Le travail doit payer le travail doit payer pour tous les Français. Les salariés verront donc leur salaire Net augmenter grâce à la suppression de leurs cotisations chômage et maladie. Les indépendants seront plus nombreuses à bénéficier des régimes simplifié d'imposition et à pouvoir tenir une comptabilité allégé. Je vous demande également. De compléter votre regard sur le PLF avec un regard sur le PLFSS présenté par la mise de la Santé, Agnès Buzyn et par le ministre de l'action et des Comptes publics Gérald Darmanin. Rehaussement du minimum vieillesse, revalorisation de la location adultes handicapés. Mesures en faveur des familles monoparentales. Plan d'accès territoriale aux soins. Nous avons fait en sorte. Que les Français les plus fragiles. Ceux qui sont touchés par le handicap, ceux qui sont touchés par la maladie. Ceux qui sont dans les situations les plus précaires. Puisse continuer à bénéficier du soutien de la nation. Ces mesures redistributives sont importantes. Et elles sont justifiées, quand elle concerne les publics qui en ont le plus besoin. Nous estimons. Et cette question des inégalités. Reste une question majeure. Et que l'on peut concilier ambition économique pour la nation. Et réduction des inégalités. Et je vais même vous dire ma conviction profonde. C'est justement en retrouvant une ambition économique pour la nation. Que nous retrouvons des marges de manoeuvre. Pour réduire réellement les inégalités. Nous retrouvons des marges de manoeuvre nationales. Mais nous retrouverons aussi une crédibilité internationale pour porter ce combat de la lutte contre les inégalités. J'ai organisé il y a 2 jours au ministère de l'économie et les finances. Une réunion avec. Les acteurs de l'économie, des chercheurs, des universitaires et présidents d'entreprises et responsables politiques. Pour ouvrir cette réflexion sur la lutte contre les inégalités face aux ruptures technologiques, comment faire en sorte. Que les ruptures technologiques ne se traduise pas par toujours plus d'inégalités entre les nations. Et à l'intérieur des nations. Comment ne pas être interpellé. Par la puissance de ces géants du numérique dont je vous parlais il y a peu de temps. Par le niveau de capitalisation jamais atteint. Par ces grandes entreprises du numérique, qui ont des niveaux de capitalisation qui se chiffrent en dizaines de milliards de dollars. Comment ne pas être interpellé par le fait que sur 7 de ces géants du numérique 5 sont américains. 2 sont chinois. Comment est-ce que l'Europe peut retrouver sa place. Dans ce combat économique : comment faire en sorte qu'il n'est pas demain quelques grandes puissances et des dizaines de nations qui perdent leur souveraineté. Leur indépendance et leur capacité à créer de la richesse, comment éviter qu'il n'y a, dans une nation ce qui gagne d'un côté. Et ceux qui perdent de l'autre. Comment éviter que les riches soient toujours plus riches et les pauvres toujours plus faible. Comment préserver la capacité d'une nation. à faire émerger une classe moyenne Mesdames et messieurs les sénateurs, ce n'est certainement pas en redistribuant l'argent que nous n'avons pas des richesses que n'avons pas créé que nous arrivons à lutter contre la pauvreté et contre les inégalités dans notre pays. Le projet de budget que nous vous présentons avec Gérald Darmanin. Vise précisément. à relever ces défis. Retrouver le chemin de la croissance. Retrouver le chemin de l'emploi. Valoriser le risque récompenser le travail, soutenir nos entrepreneurs. Retrouver la crédibilité de la parole française, en Europe et la capacité de la France, apporter sa voix dans le monde, celle de la justice et celle de la liberté, je vous remercie. Merci, merci Monsieur le ministre. Dans la discussion générale, la parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'action et des Comptes publics. Monsieur le président, Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, cher Bruno, mesdames et messieurs, sénateur, permettez-moi, comme Bruno Le Maire d'abord d'avoir un mot particulier pour votre rapporteur général général aujourd'hui saluer le sénateur Longuet et vous dire effectivement que que nos pensées les plus affectueuses et peu républicaine, la compagnie. Quelques mots pour compléter si me permet les propos de monsieur mise économie et des finances pour insister sur 4 points qui me semble-t-il, font écho au débat qu'on a déjà eu ce projet de loi de financement pour les 5 ans qui viennent, qui sortaient pas normatif mais qui nous a permis, temps lors de ce débat que dans le PLFSS on a évoqué les questions, notamment de la bascule de de souligner l'action du gouvernement en matière budgétaire, c'est 4 points seront la fin services à Sion de notre budget et les efforts que nous faisons pour le l'obtenir un point particulier en ces jours de congrès des maires de France et particulièrement de votre assemblée sur la politique en matière de collectivités locales, la transformation de notre économie et enfin le soutien au pouvoir d'achat de nos concitoyens, le 1er point sans doute le plus important pour le ministre des comptes publics et je suis, je sais que votre chambre est particulièrement attentif à la sa série station budgétaire et il y a sans doute encore beaucoup de travail à faire, vu que la marche est grande, mais enfin, je remercie le rapporteur général de l'avoir souligné lors du 1er débat que nous avons ensemble je remercie l'Assemblée nationale, de l'avoir fait également, y compris le président Woerth et personne pour Kim dans tous beaucoup de respect, j'ai Carrez, ancien président de la commission des finances remercié aussi le Haut Conseil des finances publiques et les remarques de la Commission européenne sur le fait que le budget de la nation, à essayer de combler les sincères, ils assurent les plus flagrantes que année après année, les gouvernements ont accumulé. La Cour des comptes a rendu un rapport au lendemain de la nomination du gouvernement, ce rapport souligne et 7 milliards de sous-budgétisation tant sur des questions qui relevaient des dépenses de guichet et notamment sur l'allocation adulte handicapé au sauna politique du logement, que des sur des sujets de sous-budgétisation qui qui a entaché la sincérité de notre budget, je pense notamment au ministère de l'agriculture qui a connu une dérive très important dans les années précédentes, chose est faite désormais que les 7 milliards de budgétisation tant pour l'année 2017, bien sûr que pour l'année 2018 et revenir sur ce point me paraît normal, au moment où les parlementaires et c'est bien logique, contrôle l'action du gouvernement, l'utilisation des deniers publics et doivent s'appuyer évidemment sur des chiffres qui sont les plus vraisemblables, possibles. Bien sûr, la vie n'a pris comme la vie d'une commune comme la vie, entreprise connaît des difficultés qui ne sont pas toujours prévisible dans un budget, il se pourrait que le gouvernement revienne vers vous pouvez expliciter mais il apparaît très anormal et pour le moins non respectueux du débat parlementaire, que le gouvernement n'applique pas les chiffres qu'il connaît au moment il vous parle que ce travail a été fait a été bien fait, je remercie les services mais je remercie aussi les rapporteurs, c'est assez rapporteurs spéciaux, quelles que soient leurs membres de groupes politiques pour souligner la où le gouvernement peut encore faire des efforts et je serai ouvert évidemment aux critiques lors du débat parlementaire sur cette question. Je souhaiterais d'ailleurs Monsieur le Président, que vous évoquez, avec le président de l'Arche et comme j'ai évoqué avec le président de Russie que nous puissions, revoir la procédure parlementaire. Il est évident que si le Parlement souhaite contrôler davantage l'action du gouvernement, notamment pour suivre les évolutions budgétaires encore faudrait-il que j'ai une discussion commune sur les vols recettes entre le PLFSS et le PLF, voilà que nous parlons du coût du travail d'un côté et que nous parlons du PLF, de l'autre, alors que, évidemment, pour les Français, c'est la même poche c'est les mêmes parlementaires qui contrôle le même budget gouvernemental mais également je crois qu'il faut revoir notre c'est-à-dire budgétaire de sa série station l'incroyable originalité qui consiste à voir les ministres une seule fois par an, pour parler de leur budget et de voir les rapporteurs spéciaux qu'une seule fois par an au moment de ce contrôle ne me paraît pas de bonne politique, surtout que nous allons passer quelques semaines voire quelques mois, pour ma part sur un débat budgétaire, alors nous allons passer une demi-journée d'été sur la loi de règlement, ce qui ne paraît pas être bon, ni pour le gouvernement, ni pour le parlement ni même effectivement pour la démocratie ainsi plus de temps pour le contrôle de l'action gouvernementale, un petit peu moins de temps pour le contrôle du budget peut-être plus de présence des rapporteurs, y compris lorsqu'ils appartiennent à l'opposition dans le débat budgétaire que je peux avoir avec les ministres-voilà ce que je propose à votre assemblée et donc proposé aux rapporteurs sénatoriaux de travailler plus en amont et de travailler plus en aval. En ce qui concerne la dépense publique dont nous pensons qu'elle est bien sûr parfois un bien pour notre société, mais malheureusement. Un peu grossière ces derniers temps, nous devons lutter contre son inflation. Alors nous allons essayer de tenir la promesse du 1er ministre devant son discours de politique générale de limiter cette dépense publique et si possible à 0 nous n'avons pas totalement réussi. Tant que la dépense publique, évidemment, je lisais encore ce matin un excellent éditorial dans le journal les Échos c'est difficile le terme utilisé par l'éditorialiste était drogués à la dépense publique, si nous partons du principe que cette dépense publique effectivement amène notre pays à être parfois un petit peu obèse souvent contradictoires dans la demande de gestion des deniers publics et lorsque l'on porte la main sur les économies de les refuser, nous avons la fierté nous présentait que Bruno Le Maire, un budget qui prévoit une augmentation des dépenses publiques de 0 5 C'est trop par rapport à 0 mais c'est 2 fois moins que dans les 2 dernières années précédentes et je pense que c'est un maître au courage du gouvernement. que la trop grande dépense publique fait naître la trop grande fiscalité et trop de déficits et trop effectivement de dettes, il faut diminuer la dépense publique, évidemment le faire sans mesure paramétrique avec le plus de transformation possibles pour baisser la fiscalité, ce qu'a évoqué Monsieur musée Économie, des Finances et pour baisser à la fin, notre déficit et notre dette, deuxièmement, je voudrais évoquer devant vous, c'est la question et je m'y attarderai un petit peu des collectivités locales. Dans le projet de loi que présente le gouvernement il y a une nouvelle façon d'imaginer les relations entre l'État et les collectivités locales. Bien sûr, les élus demandent que les efforts qui sont faits par leur leur propre administration locale soit désormais des efforts proportionnés à leur part dans la dépense publique. Ils ont raison, jusqu'à présent, l'État a trop demander aux collectivités locales par rapport à son propre travail. Cependant, il faut souligner que l'État a des dépenses différentes des collectivités locales et chacun le comprendra, dépenses régaliennes que non pas les collectivités locales et un quart des dépenses de l'État sont pour les collectivités locales, mais il est tout à fait vrai que le 5ème que représentent les collectivités locales dans la part de la dépense publique est aujourd'hui un 5ème qui représente plus en économie, surtout si l'on considère les années précédentes, et notamment les baisses de dotations.

La part des collectivités locales dans l'effort de la dépense publique sera d'un 6ème alors qu'elle représente un 5ème et l'État effectivement fera le plus gros de cet effort, il y a beaucoup à rattraper et il a beaucoup à changer et à transformer. Le principe est donc la contractualisation. Ne pas toucher à la quasi-intégralité des communes de France et considéré que pour toutes les communes de plus de 50000 habitants, tous les départements, toutes les régions, les 319 que nous évoquions, effectivement, il n'y a point de baisse de notation, c'est la première fois depuis 2010 mais il y a un encadrement d'une augmentation trop importante de la dépense publique, nous aurons l'occasion d'y revenir, il ne s'agit que du fonctionnement et non pas d'investissement et il s'agit bien sûr de donner également aux élus, la marge de manoeuvre nécessaire pour tenir cette marge de dépenses, ce qui veut dire revoir la façon dont les élus peuvent gérer leur masse salariale et notamment le gvt, vous constaterez que dans le projet de finance le jour de carence est rétabli et le point d'indice n'ait pas augmenté, je crois que c'est une mesure qu'attendaient les élus locaux, puisque lorsque l'État décide d'augmenter le point d'indice, souvent c'est les collectivités locales qui le paye, il nous apparaît nécessaire de réformer évidemment ce plan la réforme que nous avons des collectivités locales est réformes de confiance, pas de baisse de notation, une légère augmentation, même des dotations une délétère qui restent au même niveau que l'année dernière, qui a été opportunément augmenté, mais c'est le jeu, la veille de l'élection présidentielle et une cils qui restent identiques pourront reposer la question des variables d'ajustement qui crée la difficulté bien sûr de dotations qui sont peut-être un peu vieilli, et j'ai pris mon engagement lors de après la lecture à ce national de revenir en seconde lecture dans votre chambre comme devant la semaine nationale sur la desserte épée qui ne paraît pas être une bonne période d'ajustement, le gouvernement fera la correction sur ce point. La question la transformation a été évoqué, je voudrais souligner, indépendamment de la baisse de la fiscalité qui a évoqué le ministre de l'Économie et des Finances, lequel je ne reviendrai pas parler évidemment de la question très important de la transformation de nos politiques publiques et c'est la première fois que dans le budget de la république particulièrement ministère unique de 700 millions d'euros a été, qui a été créé 200 millions d'euros dès l'année prochaine pour permettre transformation transformation numérique, transformation des services publics, évitons peut-être des décisions un peu paramétrique dans la RGPP que la nappe a pu apporter quelques bonnes solutions en aparté, parfois des mauvaises, c'était le cas notamment dans la police nationale, ayons dans la revue des politiques publiques, émission plus intelligente pour savoir ce qu'on doit changer, ce qu'on doit renforcer et ce qu'on doit limiter en adaptant notre pays à la modalité bien sûr de la vie des collectivités locales, des entreprises et de nos concitoyens le budget que nous vous présentons prévoit 3 grandes transformations et des baisses de crédits budgétaires, c'est le cas de la politique du logement, nous en viendrons ou 40 milliards d'euros sont dépensés chaque année pour 4 millions de mal logés, malgré tout, il y a donc sans doute les transformations très importantes à faire, on aura l'occasion d'en parler longuement, me semble-t-il, c'est le cas de la politique du travail où effectivement la diminution du nombre de contrats aidés, et l'argent mis dans la formation qualifiante montre une transformation de la politique publique et c'est le cas dans la politique des transports, où nous avions tous garder des idées très important de dépenses sans comprendre que la fin de l'écotaxe a mis fin aux recettes, ce qui évidemment ne pouvait pas fonctionner, on aura l'occasion d'y revenir et cela fera écho aux Assises de la mobilité il y a des Budgets qui augmentent, même si je voudrais cigare devant votre assemblée, qui ne semble pas être un mauvais ministre et pourtant mon budget baisse comme quoi de Économie, des Finances, électeurs avec moi, ce n'est pas je dépense, donc je suis bon, c'est quelque chose d'important à souligner, et ce n'est pas parce qu'on est un budget qui baisse qu'on ait pas budget prioritaire, mais enfin il y a des dynamiques, il ne faut pas ignorer, d'abord, la dynamique de protection notre pays un budget d'augmentation de l'armée sans précédent depuis des années, du général De Gaulle, un milliard, c'est un milliard 8 chaque année pendant 5 ans, une augmentation du ministère de l'Intérieur, une augmentation du ministère de la justice, le régalien est au rendez-vous des augmentations budgétaires, une augmentation sans précédent également depuis les années 80 je souhaiterai souligner du budget de l'Éducation nationale et de l'université, c'est un point extrêmement important évidemment, c'est une priorité gouvernementale, notamment pour les universités qui font face encore cette année à 40000 emplois 40000 pardon étudiants supplémentaires, enfin un certain nombre de ministères dont les crédits n'augmente pas mais ne baisse pas et vous savez à quel point il est parfois difficile de lutter contre tendanciel je remercie chacun des membres du gouvernement qui viendront au tour à tour, vous dire à quel point ils ont été heureux de ses arbitrages et de la maîtrise de la dépense publique. Enfin, dernier point, la question du pouvoir d'achat est une question très importante qui a relevé monsieur mise Économie et des Finances, mais je voudrais revenir sur 3 : rapide, sujet qui nous intéresse, le dégrèvement sur la taxe d'habitation qui concernera 80 pourcent des Français, je me suis encore expliqué ce matin avec les maires de France, cette dégrèvement est prévu dans la loi et suffira évidemment la base de la dynamique 2 habitants de nouveaux locaux, et de ce que déciderait la commission des finances, mais il faut aussi dire qu'effectivement, et nous attendons tout ce discours du président de la République qu'un impôt qui est certes juste c'était Xabi tation et on a eu aussi beaucoup l'occasion d'en parler et tout aussi injuste, il reste 20 pourcent des contribuables qui la paye et même si, mais on l'a toujours dit, monsieur le sénateur Dallier et même si la baisse que nous vous proposons 10 milliards de baisses de fiscalité pour les concitoyens qui paieront jusqu'à 2500 euros nets de revenus par personne, voilà une bonne mesure de pouvoir d'achat pour l'instant des des classes modestes doit être revu et la fiscalité locale doit être revu, évidemment, et nous y reviendrons avec toutes les questions qui sont celles autour des valeurs locatives, il est tellement urgent de réviser leurs locatif que voilà 45 ans qu'on n'a pas fait et que Georges Pompidou, président de la République Chaban-Delmas 1er ministre c'était les valeurs locatives il tellement urgent que c'est pas locative et du a peut-être changé, que nous devons le faire dans le 6 mois qui viennent, alors que, vous comprenez bien que cela est si compliqué, d'autant plus que la valeur locative des locaux commerciaux, réforme qui a mis 7 ans à être appliqué, donc je suis le ministre qui va désormais l'appliquer sera en cette pleine dans 12 ans que nous avons une période à 20 sur 2 ans, c'est-à-dire que dans 19 ans il y aura une réforme locative alors commerciaux, tout le monde comprend bien la difficulté très forte de ne pas toucher d'une main tremblante, ce genre de fiscalité, tant qu'on ne sait pas exactement quel Fister fiscalité locale nouvelle, nous allons appliquer et que nous ferons évidemment priorité avec votre chambre et avec vous, le rôle éminent que la Constitution vous confère mais enfin la baisse de la taxe d'habitation, c'est du pouvoir d'achat pour nos concitoyens, un pouvoir d'achat extrêmement concret, la moyenne de la taxe d'habitation en France et je suis bien conscient que c'est une moyenne est de 600 euros dès l'année prochaine, c'est 200 euros de moins pour 80 pourcent des Français 200 euros de moins l'année d'après, cuisent héros lors de l'année 2020, je crois que c'est une mesure sans précédent de baisse de la fiscalité pour les classes moyennes, l'augmentation de la âge pour arriver à 900 euros par mois, augmentation sans précédent également l'allocation adulte handicapé et un minimum vieillesse qui augmentera de 100 euros par mois, et dans la chronique budgétaire est inscrit dans le projet de loi de finances que vous nous présentons voilà, Monsieur le Président, en essayant de tenir les 15 minutes que vous m'avez imposé sa série stations du budget, limitation de la dépense publique, baisse de la fiscalité, nouveau contrat avec les collectivités locales, transformation de notre pays, notamment par ses missions et pouvoir d'achat qui retrouvait c'est le projet du gouvernement mais je suis sûr que le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, et vous toutes et toutes laissé sénateurs auront à coeur d'améliorer la copie gouvernementale et nous en serons très heureux, je vous remercie. Merci et si monsieur le ministre. Et merci d'avoir respecté le temps je salue la présence du président Larché qui m'a fait le meilleur de me céder sa place ce matin et je passe la parole au président Vincent et blé quelques mots d'explication. Oui, Monsieur le Président, je souhaite informer le Sénat que la commission des finances, réunis ce matin, a décidé que dans la discussion générale, comme pour l'examen des articles notre collègue Gérard Longuet s'exprimerait en remplacement de notre rapporteur général Albéric de Montgolfier et bien sûr je m'associe au nom de tous nos collègues aux voeux de plein et rapide rétablissement notre collègue de Montgolfier qui ont déjà été exprimées merci. tous nos voeux de progrès publiquement à monsieur rapporteur général je passe donc la parole à monsieur en remplacement de Monsieur Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, oui, à cet instant, mes pensées vont pour Albéric dont je partage les convictions, ce qui rend ma tâche plus facile mais dont je ne maîtrise absolument pas le talent et la compétence et je, je, c'est-à-dire que vous me pardonnerez d'être moins moins à aise ce qui ne l'auraient été sur ce sujet du rapport général le cette année 2017, vous l'avez dit se termine dans un contexte plus favorable économie européenne se porte mieux et nous pouvons espérer une croissance de 1,7 un climat qui permettra naturellement des recettes fiscales plus élevées et nous sommes, nous avons la perspective réjouissante pour le pays, porté par cette conjoncture d'obtenir un déficit public le bal inférieur à 3 ce qui nous rassemble, c'est le budget 2018 et c'est ce budget sur lequel Albéric en qualité de rapporteur général s'exprimer Albéric Montgolfier discute pas les hypothèses de croissance même si elle a précisé dans son rapport écrit ses hypothèses de croissance sont évidemment soumises à des aléas à la hausse ou à la baisse, nous espérons, nous préférons les aléas à la hausse à la baisse alors compte tenu de ses hypothèses, on s'étonne que le gouvernement ne prévoit qu'un recul du déficit de très faible ampleur de 0,1 pourcent une sorte de statu quo après, reconnaissons-le, prise en compte de l'annulation

nous avons donc un déficit qui va atteindre 2,8 pourcent du PIB, ce qui est très supérieur à la moyenne européenne, je tiens à le rappeler bien rendu compte que nous sommes le mauvais élève de la classe européenne encore et nous avons, à un taux qui ne permet pas, contrairement à l'ensemble des autres pays européens de commencer à réduire notre ratio d'endettement de la dette par rapport au PIB alors cette faible réduction ne correspond du déficit structurel ne correspond pas à nos engagements européens et Monsieur le Ministre des rythmes Montgolfier rappelait que nous avons reçu une note de la Commission européenne, signalons les risques, les risques de déviation significative, nous sommes sous un regard attentif d'un contrôleur vigilant alors pourquoi, pourquoi ne sommes-nous dans cette situation, hé bien parce que ça c'est un bon point, vous n'avez pas choisi différer les baisses de prélèvements obligatoires, c'est pas le libéral que je suis qui vous le reprochera mais vous n'avez vous avez surtout choisi de reporter d'une façon significative la maîtrise de la dépense publique et donc l'addition des 2 aboutit à ce statu quo dans le

et on ne peut pas vous en vouloir en particulier nous approuvons le prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital, qui nous permet d'envisager de nous placer à un niveau européen satisfaisant au moment même, et les sénateurs franciliens le savent, nous sommes en compétition pour devenir une place financière attractive, les mesures qui ont été prises sont bienvenues

elles, continuent d'être et c'est son terme, matraqués et matraques et c'est la raison à travers par exemple la réduction de la prestation d'accueil jeunes enfants dans le PLFSS et c'est la raison pour laquelle me votre notre commission des finances proposera de relever le plafond du quotient familial pour enfin donner un geste positif à l'attention des familles. Le 2ème sujet de désaccord, c'est l'immobilier Albéric de Montgolfier, a présenté un rapport extrêmement documenté sur le caractère parfaitement illusoire de ce concept de rente immobilière il y a des rentes immobilières sans doute il y a des adhérent d'ailleurs dans tous les secteurs de l'économie, je ne connais d'ailleurs pas de chef d'entreprise qui ne cherche pas à organiser sa propre rente rendent sont combattus et en ce qui concerne la situation des investisseurs, vous avez fait un choix que nous soutenons, qui est de permettre à l'investissement immobilier de retrouver une certaine liberté et on souhaite profondément que cette ce geste significatif encourage les investisseurs français et les investisseurs étrangers à choisir notre pays comme lieu d'investissement, ce que vous faites sur l'immobilier méconnaît gravement l'utilité de l'immobilier dans notre pays et risque de casser en quelque sorte un petit renouveau qui se manifeste dans l'immobilier 3ème point accords la hausse de la fiscalité énergétique peut toujours raconter tout ce qu'on veut mais le rapprochement de la fiscalité du diésel et sur le l'essence va sanctionner ceux pour lesquels l'automobile est un outil de travail, ce qui est le cas de l'immense majorité de nos compatriotes qui vivent en dehors des réseaux de transports en commun et qui sont ont qui ont besoin du diésel comme outil de travail, nous avons amorcé 3D 3 des accords de danse sur un un contexte général où nous trouvons que votre budget, messieurs les ministres ne se soucie guère de la maîtrise de la dépense collective alors c'est particulièrement vrai je voudrais donner un chiffre, vous aviez l'objectif de stabiliser un objectif inédit de stabiliser la dépense publique en volume en 2018 et dans tendanciellement vous avise envisager une baisse de 20 milliards d'euros. 20 milliards de baisses d'euros cette et ce n'est pas 20 milliards de baisse c'est une hausse qui est inférieur à ce qu'elle aurait pu être de 20 milliards et cette différence tendanciel vous la réduisez à 14 milliards, ce qui montre qu'en effet dans ce budget s'il y a un grand absent, c'est la maîtrise de la dépense publique, j'ajoute que cette maîtrise de la dépense publique, vous la faites porter principalement aux collectivités locales, mais c'est un sujet d'actualité, j'aurais, je ne voudrais pas interférer sur un débat qui est organisé au Sénat, certes, mais aussi, on voudrait des mers à cet instant, les collectivités locales dont les dépenses de fonctionnement serait plafonné à plus 0 5 pourcent en 2018, ce qui est parfaitement contradictoire avec les responsabilités sociales que prennent les collectivités locales pour assurer un certain certaine certaines harmonie du fonctionnement de la société française, les collectivités locales, c'est la porte d'entrée à la vie collective, lorsque l'État est absent, les collectivités locales sont présentes ce 0 5 pourcent et ressentie par les élus locaux comme une sorte de désinvolture à l'égard de leur mission

vous l'identifiez pas et on risque de constater une situation de voeux pieux, beaucoup plus de que de réelle vérité alors alors un bon point, dernier bon point dans ce ce balayage sur la dépense publique, vous ne faites pas, vous ne réduisez les par la dépense publique comme vous auriez pu comme vous auriez dû commencer à le faire au début de ce quinquennat mais au moins le les présentations des chiffes sont plus sincères chers collègues estiment que les mesures de rebelles âge c'est-à-dire restituer de la vérité, représente 4 milliards 200 millions d'euros, ce qui montre l'ampleur de la turpitude précédente puisqu'il s'agissait de Budgets insincères, raison pour laquelle, mais je crois que c'est une une orientation que vous aviez compris et accepté en son temps, nous avions refusé le débat budgétaire en 2016 pour l'année 2017, vous avez dans vos diminution 3 missions seulement qui voient leurs dépenses diminuer de plus de 100 millions d'euros, 2 d'entre elles ont ouvert un débat, travail, emploi, vous diminuer d'un milliard et demi. ne comprend et l'on sait que les contrats aidés ne sont pas des solutions de long terme, mais vous pouvez comprendre parce que vous êtes des élus locaux que l'annonce brutale le recentrage énergique et assez immédiat de ces contrats aidés, et notamment aux collectivités locales et à la vie associative, des problèmes absolument sans solution et de la même façon, de la même façon, le milliard 700 millions que vous proposez d'économiser sur la mission cohésion des territoires et Philippe Dallier en parlerai avec plus de compétences que je n'en parlerai, je ne saurais le faire sur le logement, ouvre une crise qui, à cet instant, n'est absolument pas réglé

la masse salariale par exemple va continuer d'augmenter, alors là, les chiffres sont quand même assez cruel, le président de la République, Emmanuel Macron, lorsqu'il était candidat, avait envisagé une diminution des effectifs pour le quinquennat des fonctionnaires de l'État

c'est évidemment tout à fait en dehors des objectifs que vous étiez vous-même fixé. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, la commission des finances proposera au Sénat d'adopter dès 2 amendements concernant l'un, l'augmentation du temps de travail pour rapprocher le temps de travail, moi il y a un dans le secteur public de l'État, du 30, travail moyen dans le secteur des du secteur des salariés du secteur privé et, d'autre part de porter de 1 à 3 les jours de carence, de sorte que l'on puisse augmenter la force de travail du secteur public, mis à la disposition des missions qu'ils assument avec toujours beaucoup de bonne volonté et dévouement, enfin j'évoquerai la taxe d'habitation, j'évoquerai enfin moi j'évoque rien du tout, Albéric de Montgolfier évoque la, la, la taxe d'habitation et son jugement est clair: cette réforme est injuste et précipitée, elle est injuste parce que d'abord il n'y a pas le préalable, on vous l'avez évoqué monsieur Darmanin de la la remise en cause de la vétusté des valeurs locatives, ce qui est évidemment un serpent de mer mais puisque le monde a changé et qu'il est en marche, on aurait pu imaginer qu'il est un mouvement sur les valeurs locatives, ce mouvement est reportée aux calendes grecques, ce qui est une tradition que nous poussons devant nous depuis une cinquantaine d'années se vétusté des valeurs locatives. Injustice et absurdités, la commission des des finances et je remercie ses collaborateurs a établi ainsi par exemple que pour dans 3200 communes, c'est-à-dire 10 pourcent des communes françaises, il n'y aura que cinq contribuables par comme au maximum par commune cotisant à la taxe d'habitation et dans certaines communes, il y en aura qu'un, imaginez le climat dans la vie communale et imaginons surtout le principe d'injustice qu'entraîne cette décision et c'est la raison pour laquelle je j'ajoute, il faut quand même rappeler les les des chiffres 20 pourcent de nos compatriotes. Qui continueront de payer la taxe d'habitation paye 80 pourcent du produit de l'impôt sur le revenu il faut le savoir quoi pas quand on prend des décisions, savoir ce que l'on veut faire et ce que l'on veut encourager ceux qui investissent, qui entreprennent et ce qu'il considèrent en effet qu'être actif en économie, il rend service, globalement, la communauté, même si on général leur moteur et leur motivation est d'abord personnelle

le prendre en charge la vedette, monsieur le Ministre, vous écoutez c'était s'amusant les tours de passe-passe parce que on augmente le pouvoir d'achat d'imminentes à Xabi tation mais comme la dépendance elle des comédies, des collectivités locales ne diminue pas et que l'État devra bien la rembourser, je serais curieux de savoir qui va assurer ses 22 milliards si ce n'est le contribuable de l'État

je dois dire un mot en enfin de de de présentation sur la procédure budgétaire, je voudrais simplement dire à l'Assemblée nationale où il y a une une belle majorité composée de gens enthousiastes, passionnés, qui découvrent la vie publique qui découvrent la vie parlementaire, ben ils ont raison de la découvrir, il faut un renouveau moi c'est pas moi qui le condamnerait, j'ai été jeune aussi, mais l'OS dire simplement que certes on prend du temps, a voté le budget mais c'est le prix de la démocratie et je suis hanches heureuse de savoir qu'en effet la le débat parlementaire un débat long, minutieux difficile parce que ce sont des sommes considérables et derrière les sommes, il y a une certaine conception de la vie commune du respect mutuel du projet collectif, mais le Sénat en dehors des séances et en dehors de la parole, écrit puisque la commission des finances, a par exemple présenté 41 rapport en août 2000 personnes le ministre, si oui, si vous vous avez messieurs les Ministres, la possibilité de vous nourrir de ces rapports budgétaires pour faire évoluer, et en particulier pour reprendre en main la dépense publique, voilà en conclusion et pour revenir à ce projet de loi de finances 2018, la commission des finances vous demandera de l'adopter, sous réserve, sous réserve que soient adopté des amendements concernant les familles notre compétitivité et, par conséquent, la fiscalité de l'investissement et un peu d'un certain nombre de d'économie, dépenses qui sont certes symbolique mais qui montre que l'on peut faire bouger les lignes en matière de prélèvements publics à partir de la maîtrise de la dépense du budget de l'État.

Monsieur le président, messieurs les ministres, cher collègue, nous poursuivons une session budgétaire au cours de laquelle nous avons déjà examiné de nombreux textes, cela nous a montré les inconvénients de l'éclatement de la législation fiscale entre loi de finances et loi de financement, monsieur le ministre de l'action et des Comptes publics, vous avez raison de relancer le débat sur les conditions de l'examen des textes financiers au Parlement un débat qui était un peu au point mort depuis l'échec du projet de révision constitutionnelle de 2010, la commission des finances du Sénat jouera tout son rôle dans ce travail et nous devrons examiner aussi bien les modalités discussions des différents textes dans chaque assemblée que leur calendrier de dépôts et d'examen ainsi que l'organisation de la navette, surtout si l'idée de fusionner des parties recette des lois financières prospère, mais ce sont aussi les comportements et les pratiques qui doivent évoluer, nous devons nous mettre en situation de voter en étant toujours pleinement éclairé, ce qui suppose de recevoir les réponses aux questions que nous posons, et d'avoir du temps pour analyser les propositions du gouvernement qui arrive encore trop souvent par amendements déposés fort tardivement, aujourd'hui nous sommes saisis du projet de loi de finance de l'année, sur lequel se sont penchés toutes les commissions et en particulier les 76, rapporteur pour avis les 48 rapporteurs spéciaux dont je salue l'implication l'exécution d'une loi de finances est tributaire du contexte macro-économique dans lequel elle s'inscrit, c'est sur ce point que je voudrais formuler mais premières remarques d'abord à la nouvelle majorité bénéficie pleinement des mesures visant à redresser la compétitivité de l'économie mises en place sous le précédent quinquennat le gouvernement bénéficie d'une accélération marquée de la croissance et d'un dynamisme des recettes cette reprise tient notamment aux mesures mises en oeuvre depuis 2012 pour redresser la compétitivité enrichir la croissance en emplois, le CICE, le pacte de responsabilité ont ainsi largement contribué au Net redressement des marges des entreprises observée depuis 2013 plus de points, les efforts de modernisation du marché du travail, commencent à porter leurs fruits : le nombre de déclarations d'embauches en CDI étant désormais à son plus haut historique. Les parts de marché à l'exportation sont stabilisées après une baisse continue entre 2000 et 2012 et les projets d'investissements internationaux sont en forte hausse, plus 34 pourcent 2ème remarque pour ramener le déficit public en dessous de 3 pourcent du PIB en 2017 on peut considérer que le gouvernement s'est contenté de surfer sur la reprise, le gouvernement a dramatisé en juillet, les résultats de l'audit des finances publiques de la Cour des comptes, pour finalement mettre en 9 des mesures de régulation budgétaire d'un montant comparable aux années précédentes, car 4,2 milliards d'euros avec la taxe sur les dividendes, on a retrouvé le même schéma, le gouvernement dramatise en évoquant un scandale d'État avant déboucher sur des propositions technocratiques et bien modeste de réforme de la procédure d'élaboration de la loi, en réalité, en l'absence d'embellie conjoncturelle, la prévision de déficit public pour 2017 serait nettement supérieur au seuil de 3 pourcent du PIB, autrement dit le gouvernement, loin d'avoir pris des mesures de redressement exceptionnel, s'est contenté de surfer sur la conjoncture 3ème remarque : le gouvernement a même profité de la reprise pour relâcher l'effort de maîtrise de la dépense en 2018, au risque de nous mettre en porte-à-faux par rapport à nos engagements européens. L'an prochain, le gouvernement s'est fixé pour objectif de contenir la croissance de la dépense publique à 0 bien les 5 pourcent loin de l'objectif affiché en juillet d'une stabilité de la dépense près d'un tiers des dépenses programmées sont ainsi reportés des économies

nous allons saturé dès l'année prochaine, les marges de flexibilité que nous permet le pacte de stabilité, la gravité de cette remarque va au-delà des considérations budgétaires alors le gouvernement entend porter une réforme de la zone Euro, c'est la crédibilité de notre pays qui pourrait être atteinte, la France sera le seul grand pays de la zone Euro, dont le ratio d'endettement ne devrait pas diminuer l'an prochain, ma 4ème remarque me conduit à regarder les solutions retenues par le gouvernement pour éviter une sortie de route budgétaire, si je résume, il a choisi de différer les baisses de cotisations sociales prévues pour les classes moyennes, récupérant ainsi 4 milliards et demi d'euros plutôt que de reporter les réformes de la fiscalité du capital. Justement, au-delà du contexte macroéconomique, il faut s'intéresser au budget de l'État et à la politique fiscale, d'abord, le gouvernement ne se prive jamais chargé la précédente majorité, alors que pourtant, ce projet de budget capitalise sur des mesures qui ont été prises sous le quinquennat sur les 12,4 milliards d'euros de baisse d'impôts contenues dans ce budget 5,9, donc plus de la moitié correspondent à des mesures prises par le gouvernement précédent, par exemple, la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés est un peu revu par ce projet de loi de finances, mais son principe avait déjà été voté et c'est la mesure prise par la précédente majorité qui entrera en vigueur en 2018 ensuite en observant ce qui relève des décisions du nouveau gouvernement, la situation est si j'ose dire, ou rose, ce projet de loi de finances ne porte pas la marque du sérieux budgétaire regardons d'abord le déficit de l'État, il avait baissé sans interruption entre 2016, 2012 et 2016 pour revenir à 69,3 milliards d'euros pour 2017 et 2018, je vous donne les chiffres 2017, la situation se dégrade avec 76,9 milliards d'euros et 80 2009 milliards d'euros en 2018, je m'inquiète aussi les annonces du gouvernement consistant à sacrifier le Patrimoine de l'État pour des budgétiser le financement d'annonces aux contours flous depuis 6 mois, 2 fonds doté de 10 milliards d'euros issus en tout partis de cessions de participations ont été annoncées, sans que l'on sache si l'se substituer à l'autre, comment il devrait fonctionner et sans aucune justification de la rationalité économique et financière de sécession, ce budget montre que les relations financières entre État et collectivités territoriales doivent être repensées en profondeur la loi de programmation met en place un mécanisme novateur de contractualisation censé s'appliquer dès 2018 au 23 novembre nous ne savons toujours rien de la manière dont il va s'appliquer concrètement les collectivités vont voter leur budget sans savoir où elles devront faire des efforts, comment ils seront mesurés pour le reste, cette année, se caractérise certes par une DGF qui ne diminue pas mais les dotations d'investissement, elles sont réduites de 200 millions d'euros, en raison notamment de la très contreproductif, suppression de la réserve parlementaire la péréquation progressivement en matière de finances locales arrêtons le bricolage et, osons une réforme globale, nos impôts Directs locaux sont à bout de souffle nos compensation ne font que cristalliser les inégalités de richesse, il faut changer le logiciel surtout ce budget n'est pas le budget du pouvoir d'achat, le gouvernement met en avant les quelques mesures favorables, il propose par exemple les revalorisations exceptionnelle de la prime d'activité ou l'augmentation de l'allocation adulte handicapé, mais ces allocations fond dans le même temps l'objet de réforme de leurs paramètres qui conduisent à reprendre d'une main ce que l'autre a donné au niveau agrégé et alors que les crédits des ministères progresserait dans leur ensemble de 4,4 milliards d'euros 2 missions verraient leurs crédits baisser très fortement le logement et l'emploi à chacun ses priorités en dehors de ces 2 secteurs : le gouvernement peine à expliquer comment il va faire des économies sur la suite du quinquennat s'en remettant au processus action publique 2022 qui parviendra à n'en pas douter à identifier en moins de 6 mois les leviers d'économies qui permettront de redresser nos finances publiques en matière de fiscalité la réforme emblématique en faveur du pouvoir d'achat des ménages et la réforme de la taxe d'habitation si elle franchit l'arrêt du Conseil constitutionnel, elle bénéficiera 80 pourcent des foyers qui verront leur impôt réduit de 30 pourcent en 2018 de 100 pourcent en 2020, le gain moyen par foyer est estimé à 166 euros en 2018 mais Seguin même cumulé avec celui de la bascule des cotisations sociales sur la CSG ne sera pas forcément un gain Net, il faut le mettre en regard des autres modifications apportées au prélèvements sur les contribuables modestes et moyens ou en particulier en matière de fiscalité écologique qui va augmenter le 46 milliards d'euros d'ici 2024 compte tenu de la structure de la consommation des ménages, la convergence : essence, diésel et la nouvelle trajectoire de la contribution carbone vont surtout touché les ménages pauvres, pour lesquels les mesures de compensation chèque énergie prime à la conversion ne seront pas forcément à la hauteur des surcoûts,

la politique fiscale du gouvernement se résume donc à des gains relatifs ou inexistant pour les ménages modestes ou moyens et avec un certain et conséquent pour les contribuables les plus fortunés, nous aurons se débat au moment de la discussion des articles mais je ne pourrais que m'opposer à la création du prélèvement forfaitaire unique à la transformation de l'ISF en IFI de réformes dans la combinaison reviendra à accorder aux 100 plus gros contribuables de l'ISF, un gain moyen annuel de 1 1000000 et par personne, cela ne contribuera pas à significativement amélioré notre tissu économique puisqu'on attend de cette réforme : la création à long terme de 50000 emplois seulement soit bien peu au regard du coût de la réforme 4,5 milliards d'euros voir plus de 5 à compter de l'année suivante, qui me manqueront donc chaque année au budget de l'État, nous reviendrons sur tous ces points lors de la discussion des articles et d'émissions puisque cette année nous allons selon toute vraisemblance, examiner l'ensemble du projet de loi de finances, nous verrons que ce budget est moins celui du Nouveau Monde que celui des vieilles ficelles et c'est pourquoi avec mon groupe, je ne soutiendrai pas. monsieur le président, nous passons à la discussion de la motion tendant à opposer la question préalable en effet Monsieur Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues ont déposé une motion tendant à opposer la question préalable au texte en discussion, la parole est à Madame Éliane Assassi pour la motion et pour 10 minutes. Monsieur le président, messieurs les ministres, mes chers collègues, en préambule, je vous je voudrais au nom de mon groupe adresser tous mes voeux de bon rétablissement à monsieur le rapporteur général qui a été hospitalisé ce matin

non conformité pour qui, qui décide de cette non-conformité, bien entendu, il s'agit de la soumission aux femmes critères à libéraux qui structure l'actuelle construction européenne sécuritaire que l'on appelle les critères de Maastricht, repris par le traité de Lisbonne, ce sont ces critères, refusé par le peuple en 2005 qui place depuis des décennies maintenant la rentabilité financière au dessus de la satisfaction des besoins humains, à commencer par le droit au travail par le libre accès au service public, aujourd'hui président de la République et son gouvernement répondent avec des ailes aux exigences de la Commission européenne, projet après projet des ordonnances du travail, travail à ce budget, en passant par la loi de financement de la Sécurité sociale, de la réduction des APL calamiteuse pour le logement social de la sélection à l'université, en passant par la l'alignement institutionnel sur les desiderata bruxellois, cette politique aligne totalement sur les préceptes du traité de Lisbonne, la surenchère de la commission était donc attendue, elle servira qui peut en douter de prétexte pour enfoncer le clou de l'austérité pour accélérer la casse du service public pour passer, par exemple, un cap en privatisant des éléments clés du secteur public, d'entrée, le groupe communiste, républicain, citoyen écologiste entend afficher son désaccord total son opposition totale à ce cadre contraint à ce budget, qui devient une figure imposée selon des règles dogmatique sur lesquels nous parlementaires mais surtout nos concitoyens n'avons pas de prix. Macron a-t-il été élu pour plus austérité pour la destruction du code du travail pour la baisse des APL et l'asphyxie des collectivités territoriales et leur certes et secteur public, nous ne le pensons pas cette question préalable que j'ai l'honneur de défendre aujourd'hui expriment ce rejet global et vous, vous savez tous ici qu'elle n'abrogera pas d'autres discussions puisque nos chances d'adoption, d'après ce que je crois savoir sont quasiment du seul groupe d'opposition déclarée à la politique d'Emmanuel Macron, un éditorialiste d'un journal qui ne porte qui ne pas nos idées, qualifiant de Au bonheur des riches, nous utilisons cette procédure pour permettre à l'opposition de s'exprimer clairement et fortement oui notre groupe refusent cette loi de finances 2018 Pascaline augure d'une certaine manière à nouveau quinquennat de sacrifices et de souffrance pour nos concitoyens, sans que cela ne se traduise en plus par une amélioration durable de la situation des comptes publics et de la situation économique et sociale, cela fait tellement d'années que le chantage est ainsi pratiqué à l'endroit de nos concitoyens, qu'il en devient presque indécent de rappeler les contours de cette logique de ces politiques d'austérité qui ont tant nui à la situation, ce projet de loi de finances s'inscrit dans un système idéologique qui, comme je l'ai indiqué perdure depuis des années, mais mes chers collègues, où vivons-nous. Avez-vous bien que cela fait plus de 30 ans que les salariés de ce pays, goûte aux délices de la flexibilité de l'emploi avec une bonne trentaine de type de contrat de travail existant sur le marché, cela fait plus de 30 ans que sensible aux sirènes du MEDEF et à l'époque d'Yvon Gattaz, président du CNPF, les gouvernements, les gouvernements successifs ont estimé qu'il était temps de réduire les cotisations sociales, d'alléger les charges, ce long discours le discours convenu pour créer de l'emploi, nous en connaissons le résultat, 30 ans après les premiers textes de la loi sur les faits, la flexibilité, nous offrons à 6 millions de nos compatriotes l'insécurité de périodes de chômage entrecoupées de petits boulots de contrats à durée déterminée et autres missions d'intérim la transformation prochaine du CICE en allégement pérenne de cotisations sociales, élément du salaire sans cesse réduits depuis quelques années déjà, devrait conduire le SMIC français aux alentours du SMIC, de certains pays de l'Est européen cotisations comprises, quel progrès quelle avancée ces cadeaux au patronat offert par dizaines de milliards sans le moindre résultat en matière de politique industrielle et d'emploi doivent cesser la flexibilité de l'emploi sur la durée, l'une des causes des maux dont souffre notre économie du point de vue de la compétitivité, il faut le rappeler le chômage coûte cher à la nation, il épuise les comptes publics, alors que le licenciement est une variable d'ajustement pour satisfaire des actionnaires, oui, nous ne pouvons pas parler de ce budget, sans évoquer les choix économiques et sociaux, ce qui plombe la fine les finances publiques, c'est le maintien dans une économie de rigueur dont l'objet 1er le maintien de la rentabilité financière et la stabilité de l'État, notre ambition est radicalement opposées : pour nous, c'est l'Huma dabord, et certainement pas le bonheur des riches, la politique fiscale que vous proposez avec ce budget sert également des intérêts privés minoritaires des orateurs ne manqueront pas de relever les points saillants de ce texte, agissant de la réforme de la taille des habitations de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune des portefeuilles financiers ou de la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, ce débat est fort éloignée de la situation des 9 millions de personnes vivant aujourd'hui sous le seuil de pauvreté, mais mes chers collègues, puisque l'occasion nous en est offerte, comment ne pas pointer qu'il a suffi de l'examen d'un collectif budgétaire pour que nous remarquons qu'à peu plus de 300 grandes entreprises ou groupes générait ensemble rien moins que 1000 600 20 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit 80 pourcent du produit intérieur brut du pays et s'acquitter de 94 pourcent de l'impôt sur les sociétés, soit un peu plus de 30 milliards d'euros voilà tout est dit ou presque, dans ces 2 chiffres : 1620 milliards d'euros d'un côté et 30 milliards. D'euros de l'autre côté, c'est-à-dire que, année après année, loi de finances après loi de finances, nous avons vu croître et embellir les allégements de fiscalité des entreprises qui ont généré tant de pertes de recettes pour l'État pour les collectivités locales, il est bien possible de penser que la est la matrice de nos déficits d'aujourd'hui et que fait le gouvernement si déterminé à réformer la France, hé bien continue et même il prolonge et aggrave les travers du passé en valeur brute, l'impôt sur les sociétés, ce sont 57 milliards d'euros somme à comparer avec l'excédent brut d'exploitation des entreprises, c'est-à-dire leur profits bruts qui sont évalués à 665 milliards d'euros et dire qu'il y a encore des gens pour dire que l'économie manque de fonds pour investir ses 57 milliards vont devenir 28,5 à l'arrivée, nous avons aujourd'hui un impôt sur les sociétés qui pèse au regard du PIB ce que pèse l'impôt sur les sociétés est par le gouvernement de la République d'Irlande, nous connaissons effectivement nombre de chefs d'entreprise de PME, pour tout dire, pour qui le ressenti des choses est assez nettement différente, je les comprends, ce n'est pas pour eux que l'on a baissé, par exemple, le taux de l'impôt sur les sociétés, c'est d'abord et avant tout pour que la France devienne ce qu'elle est devenue en réalité à paradis fiscal pour les grands groupes à vocation transnationale où le gaspillage du capital ira de Pair avec les plans sociaux, de tout, de tout de même pour le cadre d'incitation à l'investissement des familles 1er de cordée, cité par le président de la République, les Bernard Arnault au château juridiquement déplacé les Marc Ladreit de Lacharrière généreux mécènes faisant quelques affaires avec les Émirats du Golfe, les pratiques les Patrick Drahi, riche des dettes que vont payer les 5000 suppressions d'emplois chez SFR à leur sujet comme d'autres le temps me manque pour évoquer le scandale inouï de l'évasion fiscale de ces 1000 milliards détournés de l'économie réelle dans le monde pour la satisfaction d'une élite réduite à quelques centaines de personnes il faut dénoncer, oui, mais maintenant il faut arranger la loi rendent illégale l'optimisation fiscale et sanctionné, il faut remettre les banques au service de l'intérêt général, proposé, comme le propose mon collègue et ami Éric Bocquet réunir d'urgence une corruption sur l'évasion fiscale car c'est pas un problème planétaire, posons la question préalable, là encore, voici des gens. Le grand patronat, les riches qui ont bénéficié de la baisse du taux marginal de l'impôt sur le revenu et qui vont tirer parti de la suppression de l'ISF et qui ont aussi ont leur temps, profiter de la réforme des données des donations, voici des gens qui vont sans effort excessif. RECAP récupérés en 2018, des sommes considérables, sans commune mesure avec l'aumône publique de la baisse de la taxe d'habitation pour les contribuables modestes et moyens qui fait vaciller les collectivités territoriales, pourtant au coeur du service public et de l'investissement public en cette semaine du congrès des maires, il faut entendent l'alerte envoyé par l'appel de Grigny sacrifier les collectivités territoriales s'est briser le pacte républicain, avec d'autres de tous horizons : nous ne laisserons pas faire, nous ne suivrons pas Emmanuel Macron le gouvernement d'Édouard Philippe dans le pari sur l'avenir qu'qui viennent d'engager avec ce premier exercice budgétaire cadeaux fiscaux consistant, mais certain en termes d'effets sur l'activité baisse de la dépense publique, aggravation de la condition des fonctionnaires, absence de réponse aux urgences de la situation sociale du pays, attaque sans précédent contre les collectivités territoriales, tout cela ne peut que justifier la dedans, l'adoption de la question préalable que nous voulons que nous soumettons à votre botte, je vous remercie. Personne ne s'étant inscrit contre la la motion, je passe la parole à la Commission, quel est l'avis de la commission des finances. Alors Alors je rapporte l'avis de la Commission, nous pouvons et nous voulons débattre, donc nous sommes hostiles. Merci et quel est l'avis du gouvernement. Défavorable. Merci, Monsieur le Ministre, il y a-t-il des explications de vote, je n'en vois pas. Elle Elle va être courte, c'est pour dire elle va être bonne voeux je je partage tout à fait l'avis de notre rapporteur général par intérim, je veux le dire et je suis étonné qu'il ait simplement pas dit la même chose, année ternir. Merci, cher collègue Monsieur Rambourg. tout d'abord parce qu'effectivement nous devons respecter le le débat parlementaire, il est quand même nécessaire dans notre démocratie que les les différents groupes puissent s'exprimer et puis je pense qu'il est aussi opportun que que les Françaises et les et les Français puissent observer la position de de ceux qui ont un double langage qui souhaitent peut-être que la France échoue et surtout qui n'ont pas su faire les réformes de transformation dans notre pays a besoin ce budget que nous allons étudier est un budget de transformation qui baisse pour la première fois depuis longtemps la fiscalité sur les ménages sur les entreprises qui va redonner du pouvoir d'achat à beaucoup de Français, je pense notamment à la réforme de la taxe d'habitation, nous aurons le temps en séance d'évoquer les nombreuses autres transformations qu'importe ce budget je vous, je vous invite, chers collègues, a rejeté cette question préalable Bercy. Merci, cher collègue, Monsieur, Kamerhe. Merci Monsieur le Président, messieurs les Ministres, je voulais dire, au nom du groupe de l'Union centriste, bien entendu, qu'au vu de l'argumentaire qui vient de motiver cette question préalable, nous ne pourrons la voter et donc nous allons également nous y opposer. Merci, chers collègue, je ne vois plus d'explications, de demandes d'explications de vote, je vais consulter le Sénat sur la question préalable opposée par monsieur Éric Bocquet et plusieurs de ses collègues, je rappelle que l'adoption de cette motion entraînerait le rejet du projet de la de finances pour 2018, en application de l'article 59 du règlement de scrutin public ordinaire et de droit, je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement est défavorable, il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement de scrutin sera ouvert dans quelques instants.

Le scrutin est ouvert.

Plus personne ne demande à voter. Le scrutin est clos Javid la secrétaire à procéder au dépouillement de scrutin.

Voici le résultat du scrutin numéro 29 sur la motion numéro 358 tendant à opposer la question préalable, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordé par les sénateurs aux groupes politiques et notifié à la présidence Nombre de votants : 343 Nombre de suffrages exprimés 343 pour l'adoption 14 contre 329 le Sénat n'a pas adopté. Nous passons à la suite de la discussion générale. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Julien Bargeton pour 7 minutes. Monsieur le Président, messieurs les Ministres, Monsieur le Président de la commission des finances monsieur rapporteur général en souhaitant un bon rétablissement Albéric de Montgolfier, chers collègues, le texte qui va occuper nos heures et nos journées n'est pas anodin mais un projet de loi de finances ne l'ai jamais vraiment ce projet de loi de finances intervient dans un contexte européen singulier qui a de quoi déconcerter le Brexit qui, comme tous les divorces n'est pas un moment heureux du projet européen les tensions en Espagne, les incertitudes sur l'avenir budgétaire de l'Italie est désormais une crise politique inédite en Allemagne, faute de majorité claire au Bundestag. Nous n'avons aucune raison de nous réjouir de cette situation, mais nous devons la garder à l'esprit lors de nos débats à venir, notre pays longtemps décrit comme frappées de fièvre hexagonale. Du fait de son instabilité institutionnelle et politique est à présent un îlot de stabilité sur un continent secoué par les frissons, car l'espoir né de l'élection du président de la République ne s'arrête pas à nos frontières et nous avons collectivement l'opportunité de contribuer au retour de la France en Europe, à cet égard l'avis de la Commission européenne nous poussent à agir, mais pas dans le sens d'une aggravation des déficits, nous aurons des débats parfois techniques mais cette chance historique est un aiguillon la stabilité politique n'est pas synonyme d'inertie, elle est au contraire une invitation à une transformation profonde de nos politiques publiques et de notre système fiscal, nous devons à présent agir à partir d'un diagnostic lucide sur l'état de nos comptes publics, ce qui a été fait par le gouvernement dès le mois de juillet sur les freins qui entravent le financement de notre économie, mais aussi un regard critique sur les résultats en deçà des attentes quotidiennes de nos concitoyens, la politique de l'emploi et la politique du logement, c'est définitivement le bon moment pour agir, les signes d'affermissement de la reprise de la croissance sont bien documentés par une c'est : il s'agit de tirer parti de ce contexte économique favorable pour réduire durablement les prélèvements obligatoires et réduire tout aussi d'agréablement certaines dépenses publiques, devenue inefficience. à l'inverse, la dépense publique n'est pas par nature mauvaise et il n'est d'ailleurs pas rare que ceux qui réclament la réduction de la fiscalité en première partie, soit les mêmes qui s'opposent aux mesures d'économie en seconde partie, à titre indicatif. Je rappelle que la dépense publique entre 2002 et 2008 avait progressé en volume de 2,1 pourcent par an et que le gouvernement s'est engagé dans la trajectoire pluriannuelle des finances publiques, un ralentissement inédit de la dépense à hauteur de 0 4 pourcent par an entre 2018 et 2022, entendons-nous bien sur la notion d'économie, car le groupe, les républicains avaient déjà aggravé de 10 milliards d'euros supplémentaires à l'Assemblée nationale, le déficit public en première partie éco, terme de du PLFSS au Sénat, vous avez creusé le déficit public de 7 milliards d'euros supplémentaires et de 5 milliards au moment du PLFR je ne doute pas de votre bonne volonté et l'amendement de suppression de l'impôt sur la fortune immobilière en est déjà un 1er témoignage à faire de même au cours de ce débat, vous nous aviez proposé la semaine dernière lors de l'examen du PLFR pour 2017 sur la taxe dividende d'utiliser le surcroît de recettes pour régler ce contentieux, nous n'avons pas entendu, mais peut-être était cela fatigue défendre une réduction de la dépense publique à ce moment-là, étonnant non, pour citer Pierre Desproges que vous avez affectionner Monsieur le ministre, je crois, je doute que cette attitude soit à la hauteur des enjeux du moment, il est vrai que le moment est un peu long, âgé de 44 ans, je n'ai vécu que 2 ans dans un pays avec des comptes publics en excédent car depuis 1975 nous sommes systématiquement dans le rouge, c'est dire, ne s'y ont pas la branche sur laquelle nous sommes collectivement si le Sénat et je le regrette, n'est plus une évidence pour nos concitoyens et nous devons être capables de leur redonner confiance dans l'action publique, je conçois que les formations politiques puissent avoir des agendas interne mais de noms ne donnons pas une image caricaturale notre assemblée ce budget et surtout les citoyens méritent mieux la première partie, que nous allons examiner fixe fiscalité et je souhaite m'y attarder un peu la stratégie fiscale du gouvernement passe d'abord par un allégement de la fiscalité pesant sur les ménages le principale mais non unique levier de cette politique et l'exonération de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des foyers à l'horizon 2020 la commission des finances a fait le choix que je ne partage pas d'ajourner ce gain de pouvoir d'achat qui profitera qui profitera en priorité aux classes moyennes, nous aurons, je pense, l'occasion d'y revenir au cours de ces débats et je ne trahis pas un secret en disant que le chef de l'État abordera ce sujet cet après-midi, le groupe la République en marche souhaite être partie prenante et force de proposition d'initiative sénatoriale visant à transformer notre fiscalité locale difficile à à piloter pour les élus et incompréhensible pour à peu près tout le monde l'exigence de transformation se retrouve également dans les mesures relatives à la fiscalité du capital, c'est le cas du prélèvement forfaitaire unique, l'objectif de la mesure n'est pas comme on l'a beaucoup entendu de faire un cadeau aux Français les plus aisés mais de faciliter le financement des entreprises, c'est le même souci qui anime la réforme très commentée de l'impôt de solidarité sur la fortune et qui est devenu un totem pour les 2 côtés de l'hémicycle, entre ceux d'une part, qui voit un moyen de contenir les inégalités de Patrimoine, oubliant au passage que nous sommes en économie ouverte et ceux d'autre part, qui souhaite la suppression totale de l'ISF, l'ISF est un impôt épouvantail qui n'est pas un matou dans un contexte de compétitivité internationale fille et néanmoins justifié car l'investissement augmente immobilier au-delà de la résidence principale, reconnaissons-le, n'est pas celui qui contribue le contribuent le plus à l'économie de la connaissance et d'innovation, que le gouvernement souhaite consolider, je suis également satisfait de voir que ce budget comporte des mesures fiscales attendues par les entreprises, nous aurons l'occasion d'en parler lors des examens lors de l'examen des articles non rattachés, notamment de l'impôt sur les sociétés à cela s'ajoute d'ailleurs : la transformation du CICE en allégements de charges à l'horizon 2019, quelques jours après la désignation d'notre capitales comme destination de l'agence bancaire européenne, la suppression de la tranche additionnelle de 20 pourcent de taxe sur les salaires, tire les conséquences de façon positive du Brexit pour la place financière de Paris, mon intervention ne peut être exhaustif, je rappellerai simplement que la politique fiscale n'est pas un jeu de Meccano lorsque la majorité sénatoriale a décidé de supprimer la hausse de la CSG L à déstabiliser l'ensemble de l'édifice, car si les textes sont distincts, la stratégie fiscale cohérente, il est très facile de se faire le défenseur de retraités en omettant de dire que non seulement l'exonération de la THA profitera mais aussi que la hausse de TVA que certains proposent frappera tous les retraités, y compris ceux qui ne sont pas concernés par la hausse de la CSG, telle n'est pas notre philosophie de l'action, clarté des choix fiscaux crédibilité des hypothèses retenues, contrôle des deniers publics, le groupe la République en marche a toutes les raisons de soutenir le PLF issu des travaux de l'Assemblée nationale, car il réconcilie l'eau et le feu de la politique fiscale française des 20 dernières années, l'eau et le feu de la politique fiscale des 20 dernières années, la solidité de notre économie et la solidarité entre les citoyens, je vous remercie. Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Éric Bocquet pour le groupe CRCE et pour 12 minutes. monsieur le président, messieurs les ministres, messieurs donc ce président de la commission des finances, rapporteur général que évidemment nous saluons très amicalement mais, chers collègues, nous entamons donc aujourd'hui l'examen du 1er projet de loi de finances 2018 élaboré par ce nouveau gouvernement, il s'agit bien évidemment de donner à l'État un budget pour l'année prochaine mais bien bien au-delà ce 1er budget fixe aussi très clairement les lignes directrices pour le quinquennat qui sous. Vous voyez donc, messieurs les Ministres, d'entrer dans la maison France. Ainsi, penchons-nous qu'il eut été fort utile de procéder à un état des lieux exhaustif de notre société et de la République. Liberté, égalité, fraternité, cette magnifique devise est aujourd'hui bien souvent contestée par la réalité de la vie quotidienne vécue par une très grande majorité de nos concitoyens. C'était pas des lieux qui était facile à faire, continue de nombreux documents disponibles pour ce faire, je pense aux rapports récents d'ONG comme Oxfam, le Secours populaire français ou, plus récemment encore, le Secours catholique, elles sont unanimes : malheureusement pour relater le constat qu'elles ont pu établir. Vous nous rétorquer aurait peut-être comme d'autres le firent Pavon vous que nous ne sommes plus à l'époque de Zola, certes, et c'est bien là où le bât blesse : les données pour 2017 sont absolument effarante pour un pays comme le nôtre, encore à ce jour 6ème puissance du monde. Nous ne pouvons pas faire l'économie de quelques chiffres. En 2016 les 10 pourcent des Français les plus riches détiennent 56 pourcent des richesses quand les 50 pourcent les plus pauvres se partagent 5

cette pauvreté qui prend racine dans notre pays, a bien évidemment des conséquences concrètes dans la vie de nos concitoyens 20 pourcent d'entre eux déclarent avoir renoncé à des soins dentaires, du fait de leur coût 12 pourcent à l'achat de lunettes ou encore 16 pourcent à une consultation chez un médecin spécialiste, le concept d'égalité des agents préambule est quelque peu mise à mal dans notre République. Car lorsqu'on porte le regard vers le haut de la pyramide, il y a les premiers de cordée, on se dit qu'effectivement il y a quelque argent dans ce bas monde, un magazine économique aux feuilles de papier glacé, publie chaque année en juillet, un numéro spécial, nous présentons le palmarès des 500 premières fortunes de France, il suffira ici de citer juste un extrait de l'éditorial du numéro de cette année. Je cite le constat saute aux yeux, à voir l'évolution du classement des 500 fortunes professionnelles depuis sa première édition du magazine en 96, le Patrimoine des ultra-riches en France a considérablement progressé depuis 2 décennies, les chiffres attestant de leur prospérité impressionne le nombre de milliardaires a explosé de 11 à 92 et au total, la valeur des 500 fortunes passer de 80 à 570 milliards multiplié par 7 le ministre, Emmanuel Macron, conseillère en janvier 2015 aux jeunes Français d'avoir envie de devenir milliardaire considérant ces chiffres, l'opération risque de prendre, me semble-t-il un peu de temps. Nous pourrions citer également à titre d'exemple, le cas de ces 3250 ménages les plus riches de France, qui ont transféré 140 milliards d'euros dans les paradis fiscaux, de par le monde, l'occasion aussi de rappeler le scandale de l'évasion fiscale régulièrement révélé de manière spectaculaire dans les médias et quand le tumulte médiatique ça pèse au bout de quelques jours, le silence fait et le scandale continue mais, chers collègues, rappelons-le, sans cesse la République perd chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros, c'est l'équivalent du déficit que vous vous apprêtez à voter mais chers collègues ce combat doit nous rassembler au-delà de nos sensibilités propres et il doit être mené sans faiblesse, sans compromission, c'est la mère des batailles au nom de la République et de la démocratie, monsieur le Ministre ne pensons pas que votre budget soit la bonne réponse au Costa que nous venons d'évoquer. Nous constatons d'abord qui s'inscrit dans la lignée des Budgets antérieurs, cela a été rappelé par Éliane Assassi enserrée dans les carcans que nous vous vous êtes donné après la RGPP la monnaie, modernisation de l'action publique le TSE, j'ai le dogme de la réduction de la dépense publique réaffirmé ce matin, comme si elle était nuisible par nature qu'elle ne contribuait pas elle aussi à la croissance et au développement aussi cette continuité se traduit-elle dans vos choix budgétaires. Nous détaillerons notre propos au cours des jours à venir dans cet hémicycle, nous voudrions évoqué aujourd'hui 3 mesures fortes de votre projet, à commencer par la suppression de la taxe d'habitation et commencé dans cette haute assemblée par ce sujet prend un sens évidemment très particulier ce sujet fluide abondamment débattue lors de la récente campagne des élections sénatoriales, tant il suscite toujours beaucoup d'inquiétudes chez les maires et les élus locaux, il y avait certainement une réforme à mener, ça ne fait aucun doute, en matière d'impôts locaux, elle ne doit pas évidemment éludé le sujet épineux de la valeur locative cette annonce démagogique, selon nous, et qu'en sera-t-il demain de la taxe foncière, nos concitoyens auront-ils à subir en conséquence des hausses des taxes locales et des tarifs des services publics locaux, cela signifie aussi à terme que seuls 20 pourcent des contribuables vont se retrouver à être les seuls à payer, certes on évoquait compensation par l'État mais les élus locaux conserve en mémoire la décision de suppression brutale unilatérale de la taxe professionnelle, il y a quelques années, qui devait aussi être compensé à l'Euro près mais vous le savez, telle ne fut pas le cas, le compte n'y est pas, que se passera-t-il après 2018 les communes seront privés à terme de 10 milliards d'euros de ressources, la taxe d'habitation représentent chacun le sait ici environ 35 pourcent des rentrées fiscales, ces préoccupations se sont largement exprimés cette semaine dans les travées du congrès des maires de France messieurs le Ministre les collectivités représentent encore plus de 70 pourcent de l'investissement public dans ce pays, et seulement 9 pourcent de la dette globale de la France, nous vous suggérons de les solliciter comme levier de sortie de crise et non comme une variable d'ajustement budgétaire, enfin, cette mesure est aussi combattu par nombres de personnes car elle est contraire à l'article 72 de la Constitution qui sanctuarise le principe de la libre administration des collectivités territoriales en leur garantissant leur autonomie financière, oui il faut une réforme de la fiscalité locale mais globale et en concertation pour ces raisons, nous proposerons la suppression de cet article 3 nous évoquerons ensuite l'article 11 celui qui met en place le prélèvement forfaitaire unique, là encore, point de nouveautés, cette disposition figurait par exemple dans les propositions de Monsieur Fillon, candidat des républicains à lors de la dernière présidentielle, elle propose une taxation unique à 30 pourcent elle a pour premières conséquences de revenir sur le principe de progressivité de la fiscalité en vigueur jusqu'à présent, il n'y aura plus ainsi de variations en fonction des revenus comme tout impôt à taux unique ce PF sera donc inégalitaire et profitera aux plus aisés, cette taxe s'appuie sur 2 sources : un taux de cotisations sociales de 17,2 pourcent et un temps forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8 ce dispositif peut donc générer une forme de pratiques d'optimisation fiscale à terme car les revenus du capital seront moins taxées, le dispositif est donc une véritable bombe à retardement pour les finances publiques qui transformera durablement une fiscalité déjà favorable aux plus aisés en une grande machine à redistribuer à l'envers nous voudrions également à cet instant évoqué l'article 12 visant à la suppression de l'ISF et à la mise en place de l'impôt sur la fortune immobilière déjà symboliquement le mot solidarité disparaît, ce qui dans le contexte d'inégalités aggravées évoquée plus haut, prend un sens très très particulier, ni Jacques Chirac ni s'y colle, Nicolas Sarkozy n'avait osé toucher à cet ISF monsieur Macron le fait, selon nous, ce n'est pas en supprimant un impôt socialement juste une lubie du MEDEF, entre guillemets, comme le disait lui-même Emmanuel Macron en 2014, de la France sera davantage attractifs mais autres temps autres moeurs, il est proposé par notre gouvernement de transformer l'ISF en IFI en sortant de l'assiette de l'ISF des valeurs mobilières, détention d'actions d'entreprises, l'obligation de PEA d'assurance-vie afin de diriger l'épargne vers les investissements productifs et aussi, nous dit-on, de dynamiser l'économie. Perte de ressources estimées par l'État à 3,2 milliards d'euros par an, l'effet combiné de cet impôt sur la fortune immobilière et du prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, aura des effets absolument hallucinant pour les bénéficiaires de ce dispositif, je veux ici me référer à la réponse faite par vos services, messieurs les Ministres au courrier que vous avez adressé notre président de la commission des finances, Vincent et blés le 26 octobre dernier le président interrogé vos services sur les conséquences de la mise en oeuvre et de l'IFI et du PS fut les éléments de réponse absolument édifiant inciteront quelques-uns avec le PSU, les 100 premiers contribuables à l'ISF gagneront chacun en moyenne 582380 euros par an pour les 1000 premiers contribuables le gain moyen liés au PSU s'élèvera à 172220 euros par an le bénéfice lié à la mise en place du pays fut apparaît aussi extrêmement concentré 44 pourcent du gain total est capté par le 1 pourcent des ménages dont le revenu est le plus élevé. Enfin, cerise sur le gâteau, dernière élément d'analyse pour les 100 premiers contribuables à l'ISF, le gain total lié aux deux réformes peut donc être estimé à environ un 1000000 et demi d'euros par an, soit un montant supérieur à l'ISF qu'ils acquittaient jusqu'à présent, symbole sidérant aussi que la sortie d'et autres lingots d'or de l'assiette de l'impôt, monsieur le Ministre, messieurs les milices, vous allez bientôt ressembler à Don Salluste dans la folie des grandeurs pour illustrer concrètement les effets d'autres propositions, citant le cas d'un PDG du CAC 40 qui a souhaité garder l'anonymat, détenteur d'un bien immobilier de 1000000 500000 euros et le 15 millions d'euros de valeurs mobilières diverses l'ISF actuel lui vaudrait un impôt de 195700 euros avec l'IFI il perdra la somme de 3900 euros, monsieur le président de la République aura du mal à se débarrasser dans ce quinquennat du sparadrap du président des riches, version 2 enfin un mot sur l'article 15 visant à la réduction de l'assiette de la taxe sur les transactions financières dans ce projet de loi de finances, il est proposé de revenir sur une des positions adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 2017 et qui élargissait l'assiette de la taxe sur les transactions financières françaises aux opérations dite intra-Day, c'est-à-dire dénouée au cours d'une même journée est considéré comme des opérations financières les plus spéculatives, cette extension du Champ de la TTF avaient été obtenus de longue lutte après 5 années d'âpres débats dans l'hémicycle, elle est censée entrer en vigueur au 1er janvier 2018 et contribuer à l'amélioration du rendement de ladite taxe, elle rapporte actuellement environ 1 milliard la taxe élargie aux opérations Intraday rapporterait entre 2 et 4 milliards chacun se souvient aussi en juin dernier, la Cour des comptes a publié un rapport à charge tirant taboulé rouge sur la TTF et sur son éventuelle extension sans doute convient-il de rappeler ici que ce sont bien les élus dans cette république qui fixe les règles et lève l'impôt pour financer l'intérêt général, on comprend bien le sens de ce signal fort dans l'industrie financière européenne, notamment après le Brexit rendre la place financière de Paris plus attractive pour les financiers, vous nous expliquer, monsieur le Ministre, qu'il faut encourager ceux qui prennent des risques qu'il faut libérer la fortune de taxes pour orienter les capitaux vers l'économie réelle, mais des lustres de vos prédécesseurs en France et ailleurs ont puisé aux mêmes sources du néolibéralisme nous pensons madame Fathia, qui dès les années 80, tenez le même discours dans les mêmes termes exactement la célèbre théorie du ruissellement que vous nous vendez aujourd'hui les premiers de cordée dans sa version 2017, bon, on apprend que beaucoup parmi eux leur richesse sous les cieux fiscaux plus cléments au bermuda Jersey ou à l'île de Man, non pas pour investir, mais pour se réfugier de l'impôt, cette théorie du ruissellement n'a jamais fait la preuve de son efficacité, en effet, alors que la distribution des dividendes tend à diminuer partout dans le monde, la France reste championne d'Europe dans ce domaine, vous avez raison, quand vous exprimer le souhait d'orienter l'argent vers l'économie réelle, mais votre méthode ne répond pas du tout à cet objectif, chacun sait pertinemment que moins de 2 pourcent des transactions financières dans le monde ont un lien avec l'économie réelle, cette loi de finances, aurait dû être l'occasion de s'attaquer frontalement à la question, criant des inégalités au nécessaire renforcement des services publics à la domination insolente des marchés financiers dans l'économie, ce n'est pas le chemin que vous avez choisi vos premières mesures montrent déjà leur nocivité, nous évoquions tout à l'heure, la grande inquiétude des élus locaux, en réaction aux annonces faites cette été sur les collectivités, ainsi, Monsieur le Ministre votre budget va aggraver les inégalités, allez vous appliquer la double peine demain aux plus démunis, allez-vous persister dans vos choix généreux à l'endroit des plus aisés, l'état des lieux évoqués initialement dans notre intervention n'est pas prise en compte, vous comprendrez dès lors que le groupe CRCE ne puisse apporter son soutien à votre projet de loi de finances 2018 merci. Collègue. La parole est à présent Monsieur Bernard Delcros pour le groupe Union centriste. Vous avez 9 minutes chers collègues.

Monsieur le président. Monsieur le ministre. Monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général chers collègues. Au moment où s'ouvre dans notre assemblée. Le débat sur le projet de loi de finances 2018. Je veux rappeler ici. Quelle sera la ligne qui sous-tendra l'action de l'Union centriste et qui guidera nos choix en toute indépendance, en toute indépendance, lors de l'examen de ce texte, comme pour les prochaines années. Notre ligne repose sur 2 idées simples. La 1ère c'est que nous devons enfin mettre un coup d'arrêt à cette sorte de fuite en avant qui nous conduit à accroître sans cesse l'endettement de notre pays, près de 2200 milliards d'euros. Au-delà même de nos engagements européens. Au-delà même de la crédibilité de la France au sein de l'Union, comme à travers le monde, il s'agit d'abord de la responsabilité que nous portons devant les générations qui viennent. Comment pouvons-nous accepter de continuer à croître sans limite la dette que nous laisserons à ces nouvelles générations. Alors bien sûr. Mettre fin à cette dérive, appel des décisions courageuses. Je pense que le moment est venu et que les conditions politiques et économiques. Peuvent être réunies pour prendre une telle orientation de façon durable. Cette décision-là. Nous les devons à nos enfants et sachez, Monsieur le Ministre, que nous serons toujours à vos côtés pour le soutenir. La 2ème. C'est que la réduction de nos déficits et de notre endettement. Ne doit en aucun cas avoir pour corollaire d'aggraver la fracture sociale et la fracture territoriale de notre pays. Avoir pour corollaire de pénaliser davantage encore les plus fragiles de nos concitoyens les plus fragiles de notre territoire. Le risque existe. Et nous le savons. Il est donc impératif d'accompagner cette politique budgétaire. 2 mesures renforcées de solidarité. Cela s'appelle tout simplement l'équité sociale et l'équité territoriale, nous le devons à nos concitoyens, nous le devons aux territoires de France. Monsieur le Ministre, vous l'aurez compris redresser la situation financière de la France, tout en veillant avec exigence, à réduire les inégalités sont nos priorités, telle est la ligne de crête le long de laquelle nous souhaitons vous accompagner. Concernant les grands équilibres de ce budget, les données macroéconomiques notre collègue Michèle Kahn être. Il reviendra et je veux pour ma part abordé plus précisément la question des collectivités locales. Tout d'abord, celui de la suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des ménages. Le candidat s'y était engagé. Le président au nord cet engagement. Tenir les engagements doit devenir une constante, si l'on veut réussir à réconcilier nos concitoyens avec l'action publique. Nous sommes favorables à un allégement des charges qui pèsent sur les familles les plus modestes, d'autant plus dans un contexte de hausse de la CSG. Je sais que sur la suppression de la taxe d'habitation, les avis sont partagés. à titre personnel, tout à fait personnel, je suis favorable à la suppression de cette taxe, qui pénalise plus particulièrement. Les Terres, les habitants des territoires les moins peuplées, pour autant, 2 questions se posent : premièrement, comment peut tant imaginer. Maintenir durablement cette taxe pour 20 pourcent des ménages alors que tout le monde s'accorde à dire qu'elle est profondément injuste. Deuxièmement. Cette mesure ne doit en aucun cas se traduire par une perte de recettes pour les collectivités locales, pas plus que par une dégradation de leur autonomie fiscale. Alors, vous avez pris en compte la réalité de ce risque et l'inquiétude des élus locaux. Et vous avez répondu par un dispositif de dégrèvement d'une part, et la possibilité pour les collectivités d'augmenter leur taux d'autre part. C'est une réponse concrète. Et positive jusqu'en 2020. Mais au-delà, le choix du dégrèvement n'apporte pas suffisamment de garanties aux élus. Alors, cette mesure ne doit-elle pas amorcer une réforme plus globale de la physique et le local, et dans ce cas-là, sur les favorable, Monsieur le Ministre a engager une concertation avec le Sénat, représentant des territoires et des collectivités et notamment via sa commission des finances, avec 2 objectifs rendent la fiscalité locale plus juste et garantir l'autonomie fiscale des collectivités dans la durée, sur la question des dotations. Les collectivités, je le dis, telle que je le pense, ne pouvait pas être absente de l'effort national de redressement des comptes publics. Elles Hyunday heure largement contribué et je rappelle qu'au terme de ces dernières années, le montant annuel de leurs DGF accuse une baisse de près de 11 milliards d'euros, 11 Désormais, il est impératif que les collectivités cancer leur marge d'action. Pour 2018, vous nous proposez un pacte global et cohérent. La fin de la baisse de la DGF. La création d'une ressource dynamique pour les régions par l'attribution d'une part de TVA. La hausse de la péréquation verticale qui s'accompagne néanmoins d'un élargissement de l'assiette des variables d'ajustement qui intègre désormais la desserte épais du bloc communal, ce qui n'est évidemment pas sans incidence sur les dotations d'un certain nombre de collectivités vous proposer le maintien de la péréquation horizontale, avec un pic stabiliser le maintien de la dotation de ce de de soutien à la messe se marrent local qui a été créé en 2016 qui subit cependant cette année une légère baisse enfin ou proposer aux plus grosses collectivités un contrat visant à limiter à plafonner la hausse de leurs dépenses de fonctionnement. Il sera important. Que cette démarche contractuelle, que nous soutenons tiennent compte des situations financières de chacune des collectivités, je pense en particulier. Incertaine départements qui doit faire face à une hausse importante des allocations individuelles de solidarité des dépenses subit sur lesquels elles n'ont pas de prise. Dans l'ensemble, Monsieur le Ministre, nous partageons les grandes lignes de vos orientations pour les collectivités, même si sur plusieurs points, nous proposerons des modifications ou des adaptations. Je veux revenir un instant sur les inquiétudes de nombreux élus, ils sont réunis en congrès, donc nous le saluons à l'occasion, je pense en particulier aux élus des plus petites communes, ils ont besoin de visibilité sur la fin de leur mandat. Entre baisse des dotations ces dernières années, incertitudes sur l'avenir et discours ambiant, ils ont besoin d'y voir clair. Je souhaite. Que vous puissiez les rassurer et leur donner de la visibilité. En leur garantissant le maintien de la DGF sur la fin de leur mandat, sur les 3 prochaines années. Monsieur le Ministre. Le texte dont nous commençons l'examen aujourd'hui. Traduit une volonté de réforme que nous approuvons. Il introduit de nouvelles mesures que nous soutiendrons. En revanche, d'autres dispositions doivent être amendé certaines entièrement examiner comme c'est par exemple le cas pour les dispositions concernant le logement. Qui ne répondent pas aux enjeux de l'habitat. Qui ne sont pas suffisamment équilibré et qui pénalise par ailleurs les territoires ruraux nous contribuerons donc activement au débat budgétaire qui s'ouvrent, soyez assuré que l'Union centriste sera un partenaire exigeants et attentifs à vos côtés pour réussir à répondre aux enjeux de notre pays, je vous remercie. Merci, cher collègue. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Emmanuel Capus. Pour le groupe, les indépendants et pour 6 minutes.

Monsieur le président, Monsieur le Ministre, Monsieur le président de la commission des finances Monsieur le remplaçant du rapporteur général, mes chers collègues. Nous allons débattre du 1er budget du quinquennat du président de la République, c'est donc un moment politique fort. Un moment de dialogue entre l'exécutif et la représentation nationale. Nous espérons qu'il sera l'occasion d'une discussion franche et pragmatique, avec un solide, l'intérêt général et pas les postures. Nous abordons un texte qui a déjà été abondamment commentée. Il a déjà fait l'objet de critiques, voire même de caricature, voire même d'annonces martiales de la part des uns et des autres. Certains fustigent un budget pour les riches. Oubliant au passage où nous a mené la frénésie fiscale du précédent quinquennat comme si le régime de fiscalité punitive duquel nous sortons avait fait la preuve de son efficacité et de sa capacité à relancer la croissance. Non. Nous saluons au contraire un budget équilibré qui restaure en partie l'attractivité de notre pays, relancer l'investissement dans l'économie réelle et rend du pouvoir d'achat à ceux qui en ont le plus besoin. Le prélèvement forfaitaire unique est en ce sens une bonne mesure qui nous permet de nous rapprocher du niveau européen de prélèvements sur le capital. D'autres critiquent la sincérité de ce texte. Oubliant que nous sortons d'une aire d'insincérité et d'irresponsabilité budgétaire sans précédent, dont les conséquences, hélas, ce sont eux encore sentir aujourd'hui nous nous saluons au contraire un budget qui est probablement l'un des plus sincères depuis 10 ans tant dans ces hypothèses macro- que dans les évaluations des dotations budgétaires. D'autres enfin se croit autorisé à donner des leçons de courage politique, oubliant tout au passage les renoncements du passé. à la tiédeur du pouvoir succède soudain le jusqu'au boutisme de l'opposition. Nous nous saluons au contraire un budget courageux qui ose aborder de front les grandes questions fiscales et apporte des solutions bien sûr imparfaite à de vieux problèmes français, M. le Président, je suis, je souligne justement un des points, madame la présidente, je suis légèrement points que vous avez vous-même souligné certains gouvernements de droite qui ont été cités n'ont pas été fait les mesures qui sont aujourd'hui proposées, moi j'étais à Angers, je n'étais pas encore élu Madame la sénatrice à cet égard nous voyons d'un bon oeil la suppression des 3 quarts de l'ISF, ce qu'aucun des gouvernements précédents, n'a eu le courage de faire depuis sa création, nous veillerons néanmoins à ce que le nouvel impôt sur la fortune immobilière remplissent bien sa mission qui est la réorientation de l'épargne vers les investissements productifs et qu'il ne pénalise pas à outrance l'investissement immobilier. Le groupe, les indépendants républiques et territoires estime ainsi que plusieurs mesures de ce PLF vont dans le bon sens, je voudrais néanmoins évoqué plusieurs points négatifs ou de vigilance qui appelleront des propositions de notre part au cours des débats premièrement les efforts budgétaires consentis, qui sont réelles, ne doivent pas nous tromper le gouvernement profite de la reprise pour passer sous silence un effort structurel Faible et une hausse de la dépense publique qui demeure inquiétante, les alertes récentes de la Commission européenne, révèle que la stratégie du gouvernement de reporter les efforts sur la fin du quinquennat pourrait mettre en péril nos engagements européens, nous émettons des doutes sur la soutenabilité des objectifs annoncés et sur les moyens mis en place pour les respecter, à cet égard le plan action publique 2022 apparaît modeste en comparaison des efforts que l'État devra consentir, nous sommes également préoccupés par le sort réservé aux collectivités territoriales dans ce texte, les maires que nous recevons cette semaine, notamment au Sénat sont les piliers de la République, avec les autres échelons locaux, il contribue à la vitalité de notre démocratie et à la qualité de nos services publics. Nous veillerons à ce que la refondation de la fiscalité locale que nous savons tous nécessaire ne se fasse pas au détriment de leur liberté et de leur capacité d'action. Nous ferons des propositions pour que la suppression de la taxe d'habitation pour 80 pourcent des ménages français ne se traduisent pas par une perte d'autonomie financière pour les communes, nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réforme d'ampleur des valeurs locatives qui sont obsolètes et injuste, mais il nous semble qu'on prend trop souvent ce serpent de mer comme prétexte à l'inaction, la mesure du gouvernement imparfaite est perfectible, a le mérite de poser les bonnes questions. C'est peut-être en effet le plus grand mérite de ce projet de loi de finances, il pose de vraies questions de société et prépare l'avenir après de nombreuses années de faux-semblants. De renoncement ou de facilité. Dans ces conditions, un esprit d'opposition systématique pourrait nous faire manquer collectivement un rendez-vous avec la transformation du pays. Pour cette raison le groupe les indépendants républiques et territoires est prêt, messieurs les Ministres, à travailler avec vous pour améliorer ce texte, nous le ferons en responsabilité, mais sans complaisance, avec la volonté d'agir au service de l'intérêt national. Merci, cher collègue dans la dans la suite de la discussion générale, la parole est à monsieur Stéphane Ravier pour les non inscrits, vous avez 5 minutes chers collègues. Monsieur le Président, messieurs les Ministres, monsieur le ministre, monsieur général que je souhaite à mon tour les voeux de prompt rétablissement, mes chers collègues, je ne tournerai pas autour du pot, le Marseillais, que je suis ira droit au but : votre projet de loi de finances est en opposition complète avec notre vision de philosophique et politique de la société française, il s'inscrit dans la continuité avec ce que vos prédécesseurs ont infligées à nos compatriotes depuis des décennies, tout d'abord, votre budget est résolument en tournée vers les plus riches, abandonnant à leur sort les classes moyennes, que ce soit clair : je ne suis pas de ceux qui compartimenter, diviser les Français, en les enfermant dans des cases ou dans des classes, je laisse à d'autres le soin de le faire, je sais qu'ils sont nombreux, les volontaires à vouloir diviser les Français, y compris dans cet hémicycle, mais force est de constater que votre politique s'attaque aux classes moyennes, alors qu'elle caresse dans le sens du poil, les grandes puissances financières ultralibérale et déraciné remplaçant lien Yacef par un impôt sur la fortune immobilière, le gouvernement fait la part belle aux placements financiers au détriment de ceux qui détiennent un ou plusieurs biens immobiliers, la volonté de privilégier la détention de valeurs boursières au détriment des biens immobiliers mettent ainsi à nouveau en lumière la philosophie politique d'Emmanuel Macron partout : il faut détruire les attacher les Liens et s'en prendre à la France, durable, qui est aussi la France des propriétaires, la finance n'est pas l'ennemi de l'Élysée, elle ne l'a d'ailleurs jamais été quitte à envisager une réforme de l'ISF, la formule la plus juste serait à l'inverse, de mettre en place l'exonération de la résidence principale, une mesure favorable aux contribuables assujettis à l'ISF, essentiellement à cause de la valeur de leur Patrimoine immobilier fruit souvent d'un héritage familial ou d'une vie de labeur, le maintien de ce Patrimoine paraît vital pour notre pays, à l'heure du grand déracinement, c'est toujours cette même philosophie que vous qui vous anime, avec l'instauration de votre prélèvement forfaitaire unique de 30 pourcent sur les biens immobiliers sur les biens vous choisissez non seulement de ne pas lutter contre l'immigration de masse, mais de la favoriser un augmentant le budget de l'aide médicale d'État et un augmentant celui dédié à l'accueil des migrants, monsieur Macron a beau communiqué la réalité de votre budget annonce urbi et d'orbi que la France continuera à accueillir toute la misère du monde, vous choisissez toujours plus, Union européenne, en augmentant le de plus de 2 milliards d'euros, la contribution de la France à ces institutions vous étrangler toujours plus les collectivités locales en supprimant la taxe d'habitation et en abaissant la dotation globale de fonctionnement des collectivités ou fermer les yeux sur les vrais problèmes qui polluent nos banlieues et nos quartiers, la politique d'immigration massive, l'insécurité, le communautarisme, la haine de la police et de tout ce qui peut représenter la France et l'État et vous mentez et vous maintenez coûte que coûte une politique de la ville de ruines dans l'inefficacité a pourtant été maintes fois dénoncée par la Cour des comptes, pendant ce temps, les classes moyennes et les Français les plus modestes trinquent, augmentation du prix du diésel du tabac des péages, des compagnies d'autoroutes à qui vous avez bradé notre réseau et bientôt viendra le 1er janvier avec ce que l'on n'ose encore présenté comme étant les traditionnelles augmentations et pour quel résultat une Union européenne qui pour il était littéralement le quotidien nos compatriotes avec d'énormes infernal quant à l'armée, si le budget annoncé ce serait sans précédent, il reste largement en deçà des besoins réels et urgent pour que notre armée puisse mener ses missions à bien maintenant, vous me permettrez monsieur le ministre, monsieur le président, mes chers collègues, cette petite indiquerait digression, pour revenir sur un événement survenu la semaine dernière lors de notre lors de notre examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale, alors que j'ai présenté est proposé 2 amendements visant respectivement réserver les allocations familiales aux familles françaises dont dont on au moins un parent et français et à supprimer les allocations aux familles dont un des membres a été condamné pour terrorisme notre collègue Alain Milon, membre des Républicains mais dont le coeur est en marche, a pris la parole pour exprimer son étonnement et saisir la présidence, je le cite je le cycle qui ces amendements écrit me semble discriminatoire et je me demande comment ils sont arrivés jusqu'ici, je tiens à condamner de la manière la plus ferme que ce qu'il qu'il soit, cet appel à la censure, il y a vous interpellez, vous tous, mes chers collègues, même vous Madame Assassi, qu'en est-il de la liberté d'expression, c'est vrai, ce n'est pas votre priorité car, est-il de la liberté d'expression dans ce pays, et plus particulièrement dans cet hémicycle qu'une voix discordante s'expriment et s'opposent dans ce lieu soi-disant du débat démocratique, on doit ne pas avoir la même opinion, mais on peut, on doit pouvoir exprimer sans être victime de la censure, nous ne sommes pas encore à Pyongyang et Alavoine Madame Madame Assassi souffrait d'entendre que 11 millions de Lecteurs puissent exprimer ici par mon intermédiaire, sur 925 parlementaires, députés et sénateurs confondus, 10 seulement représente le Front National aussi et permettez-moi de conclure, j'en appelle à la voix et la raison de l'honnêteté intellectuelle, argument contre argument, projet contre projet, projet de société contre projet de société et ce sont les Français, seul souverain dans ce pays qui décideront et pas un Fouquier-Tinville ou d'opérette, face à la situation dans laquelle se trouve notre pays face à la guerre que le terrorisme islamique lui a déclaré : nous estimons, nous, au Front national, que la France va retrouver sa place dans le concert des nations libres que notre économie dans se tourner plus particulièrement vers les classes moyennes et les plus modestes que la fracture entre nos métropole et nos arrière-pays doit être réduite sur le projet de loi de finances et mauvais, nous le pensons, nous le disons, si toutefois monsieur Milan et Madame Assassi le permettent. Merci, cher collègue, la parole est à présent à monsieur Yvon Collin pour le groupe RDSE et pour 6 minutes chers collègues. Monsieur le président, s'il vous plaît, merci, merci Monsieur le Président, messieurs les ministres, monsieur le président de la commission des finances, une pensée pour l'entrée, rapporteur général et je salue Gérard Longuet, mes chers collègues, no examinant ce projet de loi finale ce pour 2018 dans un contexte Dembélé économique, ce qui marque un changement par rapport à ces dernières années une croissance atone en particulier entre 2012 et 2013, c'est à l'évidence, une bonne nouvelle qui permet au gouvernement de fonder son son budget sur des hypothèses de croissance réaliste,

comme on les aime, au Sénat, le Haut Conseil des finances publiques relève aussi un scénario gouvernemental, je cite, prudent pour 2017 et raisonnable à 2 pour 2018, pour ma part je souscris à cet effort de sincérité budgétaire car nous sommes pas à l'abri de navire, nous le voyons malheureusement avait le fiasco de la taxe sur les 3 pourcent de dividende, si la France profite de la bonne santé de la zone Euro, on peut reconnaître aussi que certaines des mesures du précédent quinquennat portent leurs fruits, je citerai le CICE qui, malgré ses défauts, a permis aux entreprises de reconstituer leurs marges et de reprendre leurs investissements dans ces conditions, que peut on attendre du budget de l'État de l'audace de la justice et de l'efficacité sans doute de l'audace, tout d'abord clairement pour ce 1er projet de loi de finale sur la majorité actuelle, je constate qu'il n'y a rien de révolutionnaire en retrouve des recettes anciennes qui consiste à aménager toiletter aura voté ce qui conduit à une maîtrise des dépenses, certes encore insuffisant, en effet, si on peut se féliciter d'un retour à terme déficit sous la barre des 3 pourcent l'ajustement structurel ne sera que de 0 prélèvement à la source est reporté mais on a pas qu'en dehors des principales mesures, comme la création de l'impôt sur la fortune immobilière et le prélèvement forfaitaire unique l'audace a surtout consisté à instaurer un dégrèvement de la taxe d'habitation, mais sur ce point comme on peut l'imaginer, monsieur les ministres se serait bien passé de cette réforme. Nous sommes en pleine congrès des maires, et vous savez combien les efforts qui sont sans cesse demander aux collectivités locales ont dépassé la limite du supportable à travers de nombreux autres dispositifs, c'est le principe d'autonomie fiscale des collectivités locales, qui est de plus en plus affecter aussi les maires attendent d'être rassurés et j'espère que le président de la République prendra cet après-midi, Porte de Versailles, des engagements pour ne pas décevoir nos élus qui sont confrontés à en quotidien local de plus en plus difficile et nous aurons l'occasion sans doute d'en reparler dans au cours des prochains débats

de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et bien sûr à la baisse des cotisations salariales, je m'inquiète toutefois monsieur les ministres de la fin des contrats aidés qui constituent une opportunité d'embauche pour les plus fragiles, en fait, s'agissant de l'efficacité de ce budget, l'avenir nous le dira clairement le projet de loi de finances pour 2018, notamment avec les 2 dispositifs phares que j'évoquais tout à l'heure l'IFI et le pays fut vise à encourager l'activité économique, c'est un signe fort en direction des entreprises si que l'on peut toujours, bien sûr, critiquer les contours de ce de cette réforme, ces mesures comme on l'a fait pour le CICE, mais on ne peut pas ne niez espérer sans doute qu'une partie des revenus de l'épargne libéré sera réinjecté dans l'économie productive, je regrette toutefois que l'agriculture soit souvent oubliés dans les mesures d'encouragement à l'activité, alors que ce secteur en particulier l'élevage a connu une grave crise des prix ces dernières années, mon groupe sur ce point à déposer quelques amendements pour une meilleure prise en compte des besoins de l'agriculture notamment une proposition sur le micro bénéfices agricoles mais, chers collègues, comme nous sommes nombreux à le répéter chaque année notre pays doit retrouver une trajectoire à celle de ses finances publiques, c'est une question de survie dans une compétition mondiale de plus en plus difficile et contre la majorité des membres du RDSE regarde ce budget avec bienveillance et devrait l'approuver, mais nous serons bien sûr attentif aux discussions de ces procès, un jour, je vous remercie, mes chers collègues de votre attention à cette heure tardive. Merci, chers collègues, je vais suspendre la séance, elle sera reprise à 15 heures pour les questions d'actualité au gouvernement, puis à 16 heures et quart pour la suite de la discussion générale du projet de loi de finances pour 2018, la séance est suspendue.